pas provoqué la moindre réaction. Nous nous en étonnons, d'autant qu'il semblerait que nous nous dirigions dorénavant vers un débat de politique générale mercredi à l'Assemblée nationale et jeudi au Sénat.

L'exercice 2019 constituera une année charnière pour notre politique d'aide publique au développement : les décisions prises cette année détermineront si notre pays respectera l'objectif posé par le Président de la République d'une aide représentant 0,55 de notre revenu national brut, ou RNB, en 2022. En effet, étant donné le décalage entre l'engagement des crédits et leur décaissement effectif,

C'est donc à l'aune de cet objectif que nous avons analysé la présente mission, en nous demandant, monsieur le ministre, si les moyens engagés nous placent sur la bonne trajectoire en attendant la loi de programmation dont devrait intervenir en 2019 et qui détaillera les moyens consacrés à cette politique dans les années ultérieures. Tout d'abord, quelle est l'évolution des moyens financiers affectés au développement en 2019 ? Je ne m'attarderai pas sur les éléments techniques qui figurent dans le rapport spécial, mais je souligne que les circuits de financement connaissent cette année deux changements significatifs

d'autre part, le Gouvernement a choisi de « rebudgétiser » la part de la taxe sur les transactions financières affectée à l'AFD. Cette rebudgétisation a été critiquée par certaines ONG, mais nous ne partageons pas cette vision. La taxe sur les transactions financières, ou TTF, est affectée au Fonds de solidarité pour le développement, le FSD, et à l'AFD. La part affectée au FSD ne diminue pas d'un euro, et les moyens de l'AFD sont augmentés dans des proportions quatre fois supérieures à la perte de la TTF. Aussi, ces critiques nous semblent focalisées sur l'outil plutôt que sur le niveau des moyens. En définitive, en tenant compte de ces évolutions des circuits de financements, nous constatons un effort substantiel en faveur du développement en 2019, en autorisations d'engagement du moins. Au total, celles-ci augmentent de 1,4 milliard d'euros par rapport à 2018. L'effort est moindre en crédits de paiement, qui augmentent de 127 millions d'euros sur l'ensemble de la mission. Il est normal de constater un écart significatif,

Cependant, concrètement, si les moyens pour engager des projets sont là, une grande partie de l'effort financier, vous le savez bien, monsieur le ministre, est reporté aux années ultérieures. Cet effort financier est d'autant plus nécessaire que nous ne respectons toujours pas nos engagements internationaux et que nous sommes distancés par nos voisins.

et le Royaume-Uni, dont l'aide représente respectivement le double et 60 % de plus que la nôtre. Cet écart s'explique notamment par le niveau des dons bilatéraux, trois fois supérieur chez nos voisins. Sommes-nous sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 2022 ? Le budget pour 2019 n'apporte pas les réponses attendues. Le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, le CICID, a défini en février dernier une trajectoire en pourcentage du RNB, mais sans la traduire budgétairement. Notre aide publique au développement, au sens de l'OCDE, devra augmenter en 2022 de 5 milliards d'euros par rapport à 2017, sans que cela signifie qu'il faille réaliser un effort financier de cet ordre, compte tenu de l'effet de levier des prêts. Nous n'avons pas obtenu plus de précisions sur le montant des crédits budgétaires qui seront nécessaires pour y parvenir. Cette trajectoire sera définie- ou du moins il faudra y veiller -dans la future loi de programmation de l'aide publique au développement, qui devrait être examinée au Parlement au premier semestre de 2019. Des arbitrages budgétaires difficiles

Malgré ces points à préciser, nous constatons suffisamment d'éléments positifs pour accorder une confiance, certes vigilante, au Gouvernement et considérer que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l'objectif. En effet, ce budget porte une hausse inédite des moyens financiers. De même, nous observons un engagement personnel du Président de la République sur ce sujet, qu'il aborde régulièrement lors de ses déplacements et qui s'est illustré dans la création d'un « conseil de développement en prie, monsieur le rapporteur spécial. Quels sont les moyens dont disposera l'AFD en 2019 ? Ces moyens vont considérablement augmenter. S'agissant des dons, l'AFD disposera de près d'un milliard d'euros supplémentaires en autorisations d'engagement.

Concernant les prêts, l'AFD bénéficiera de 500 millions d'euros supplémentaires de bonification, qui devraient lui permettre d'accorder 1,5 milliard d'euros d'engagements supplémentaires. Par ailleurs, l'augmentation de l'activité de l'Agence remet à l'ordre du jour un sujet régulièrement abordé devant la commission : le niveau des fonds propres de l'Agence. Comme vous le savez, l'AFD est une société de financement, soumise au respect des ratios prudentiels, qui peuvent l'empêcher de prêter à certains États, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, par exemple au Maroc ou en Colombie. L'article 71 du présent projet de loi de finances prévoit une solution à court terme : l'État apportera une garantie explicite à certains prêts souverains accordés par l'Agence, et ce dans la limite de 750 millions d'euros. Par ailleurs, à compter de 2020, il faudra envisager un renforcement des fonds propres de l'agence. Par ailleurs, une des conditions essentielles de l'atteinte de l'objectif réside dans la capacité de l'AFD à absorber cette hausse de son activité. D'après les informations que nous avons recueillies, pour respecter l'objectif de 0,55 % en 2022, il faudra, à cette date, que les engagements de l'Agence s'élèvent à 17,6 milliards d'euros, soit une multiplication par deux en six ans. Demander à un opérateur de multiplier par deux son activité en aussi peu de temps n'est pas anodin, c'est donc l'une de nos préoccupations. S'y ajoutent des inquiétudes sur la capacité des pays en développement à absorber des volumes de prêts en hausse importante. un mot sur la répartition entre l'aide bilatérale et multilatérale. Le budget pour 2019 met l'accent sur la hausse de notre aide bilatérale, à travers les ressources de l'AFD. En effet, le CICID a décidé que l'aide bilatérale bénéficiera des deux tiers de l'augmentation des crédits d'ici à 2022. Cette priorité en 2019 est d'autant plus logique que l'aide bilatérale est plus longue à mettre en oeuvre que l'aide multilatérale. Nous soulignons cependant la nécessité de ne pas négliger notre aide multilatérale, dans un monde où le multilatéralisme est fortement contesté, notamment aux États-Unis. Je terminerai mon intervention en présentant l'article 72, rattaché à la mission. Cet article autorise à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de la Société financière internationale. Ces deux institutions multilatérales appartiennent au groupe de la Banque mondiale. La première intervient auprès des pays à revenu intermédiaire et dans des pays plus pauvres, à condition qu'ils soient solvables ; la seconde intervient pour sa part dans les pays en développement, mais exclusivement auprès du secteur privé.

Cette augmentation de capital s'accompagne d'évolutions au sein de la Banque mondiale conformes aux souhaits de la France, y compris en ce qui concerne sa gestion. De plus, cela permettra de maintenir la place de notre pays au sein de l'actionnariat de cette institution. de l'ensemble des éléments que j'ai présentés, la commission des finances vous invite à adopter les crédits de la mission et du compte de concours financiers, ainsi que l'article 72

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, on doit se féliciter de l'ambition de porter à 0,55 % du RNB l'aide publique au développement française. Il s'agit d'un instrument important pour lutter contre les désordres du monde : pauvreté, conflits, mouvements de population subis. Le milliard d'euros supplémentaire d'autorisations d'engagement en dons prévu pour 2019 devrait donc aider à orienter davantage notre aide vers les pays les plus pauvres, ce que nous demandions depuis longtemps. C'est pourquoi notre commission a donné un avis favorable aux crédits inscrits au sein du projet conformément aux priorités affichées par le Président de la République lui-même, si l'aide au développement, c'est mettre plus de moyens en direction des pays qui demandent plus, c'est aussi s'assurer de l'efficacité de l'aide apportée. On ne peut mesurer le succès d'une politique publique à sa seule capacité à dépenser davantage, surtout quand on peut s'interroger sur la définition de la stratégie, ses objectifs, ainsi que sur son pilotage politique et son évaluation. Ainsi, on ne peut que souscrire à l'excellent constat du député Hervé Berville et au récent rapport de la Cour des comptes à ce sujet. Concernant la stratégie, le comité interministériel de la coopération internationale et du développement s'est réuni en février dernier, après plus d'un an sans réunion. En vingt ans, monsieur le ministre, il n'aura été réuni que onze fois. Quant au conseil du développement auprès du Président de la République et au conseil d'orientation stratégique de l'AFD dont on doit se féliciter, on ne peut pas leur demander plus que de fixer les grandes orientations. Ainsi, aujourd'hui, entre la lutte contre la pauvreté et la transition écologique, entre l'aide à l'Afrique subsaharienne et les prêts à la Chine, entre la stabilisation des zones de conflit et la réduction des migrations subies, notre aide vise à atteindre des objectifs nombreux, peut-être même contradictoires dans certains cas, en tout cas peu lisibles pour nos concitoyens. Dès lors, il nous paraît difficile de faire l'économie d'un vrai pilotage ministériel, s'agissant d'une politique qui va peser plus de 15 milliards d'euros en 2022. L'Agence française de développement, qui va passer à près de 18 milliards d'euros d'engagements en 2022, a profité du retrait relatif de l'État pour acquérir une large autonomie. Si l'on veut répondre à l'ambition politique affichée, il est nécessaire que le Gouvernement et le Parlement puissent être davantage impliqués. L'aide au développement ne peut pas consister en une accumulation de projets, mais en une vraie politique de la France pour soutenir la volonté de développement des pays aidés. Vous avez compris, monsieur le ministre, l'importance que nous accordons à la préparation de la prochaine loi d'orientation et de programmation. En dernier lieu, il va de soi que le déficit de transparence et de « redevabilité » récemment relevé, de même que la trop faible part des crédits dépensée et évaluée, ne sont pas acceptables.

comme mon collègue rapporteur pour avis Jean-Pierre Vial, je me félicite de l'augmentation des moyens consacrés à l'aide publique au développement, mais surtout du choix de privilégier l'instrument des dons et le bilatéral dans la progression à venir. Une telle orientation permettra au Gouvernement d'avoir une meilleure maîtrise de nos financements et de les diriger davantage vers les pays les plus pauvres, en particulier ceux d'Afrique subsaharienne, où se concentrent pour une large part les enjeux de l'avenir. La progression des crédits se traduira notamment par une forte augmentation des moyens de l'Agence française de développement, dont les engagements devraient passer de 11 milliards d'euros en 2018 à près de 18 milliards d'euros en 2022. C'est considérable, d'autant que cette augmentation doit avoir lieu dans un contexte de moindre capacité à emprunter de certains pays émergents et, surtout, de nombreux pays africains, qui ont parfois contracté des emprunts massifs auprès de banques chinoises, avec les effets que l'on sait. Augmenter ses engagements sans diminuer en rien ses exigences en matière financière, environnementale et sociale, c'est un défi de taille qui attend l'AFD pour les prochaines années. Je souhaiterais par ailleurs souligner l'importance de la contribution française à la lutte contre le changement climatique, avec notamment un financement à destination du Fonds vert pour le climat de 775 millions d'euros sur la période 2015-2018. Cet enjeu, tout comme celui de la préservation de la biodiversité, ne peut plus être séparé de l'enjeu du développement. J'ajouterai deux remarques sur ce point. D'abord, le Fonds vert a actuellement beaucoup de mal à décaisser ses financements, et ses procédures sont très longues. Il faudra donc réfléchir l'année prochaine, dans le cadre des discussions du G7 à Biarritz, à une amélioration de sa gouvernance et de ses procédures. Deuxième remarque : nos contributions aux divers fonds climatiques ou, plus largement, en faveur du développement durable sont aujourd'hui très complexes, pour ne pas dire illisibles. Ce problème concerne d'ailleurs en réalité l'ensemble de l'aide publique au développement française. Les vecteurs budgétaires et non budgétaires sont si nombreux est très difficile, parfois impossible, de savoir précisément lesquels de nos financements contribuent à cette cible des 0,55 % que nous sommes censés atteindre en 2022, et dans quelle proportion. Des évolutions

affectée à l'aide au développement diminue en raison de la rebudgétisation des 270 millions d'euros auparavant directement affectés à l'AFD. Cette évolution, et surtout l'absence de réelle visibilité sur la trajectoire censée nous permettre d'atteindre les 0,55 % du RNB consacrés à l'aide

les moyens et, surtout, les mécanismes de contrôle qui permettront de donner un nouvel élan à notre politique de développement. Nous pourrons ainsi rejoindre les leaders européens que sont le Royaume-Uni, les pays nordiques et l'Allemagne, car ils ont déjà compris que l'aide au développement constituait un investissement indispensable, à la fois pour préserver leur influence et pour

en matière d'aide publique au développement vont donc s'accroître de manière très sensible de plus de 1,4 milliard d'euros supplémentaires. Nous nous en réjouissons, en espérant que la trajectoire budgétaire des années prochaines suivra le même rythme. nous nous réjouissons plus particulièrement que le Gouvernement ait d'ores et déjà décidé d'affecter les deux tiers de la progression des crédits de l'aide publique au développement à des financements bilatéraux, comme l'ont rappelé nos rapporteurs. rapporteurs. Ne nous méprenons pas : les financements multilatéraux ont souvent permis des avancées importantes et, à condition d'y exercer une influence à la hauteur de nos contributions, ils peuvent constituer des leviers pour atteindre nos objectifs. Ainsi, le Partenariat mondial pour l'éducation cofinance notre priorité éducative au Sahel. L'augmentation annoncée de notre contribution à ce fonds, qui a montré son efficacité, est évidemment un point positif- nous la réclamions d'ailleurs depuis plusieurs années. j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec vous, monsieur le ministre, est-ce vraiment le cas des 50 contributions multilatérales de la mission « Aide publique au développement

leur fondement et leur utilité, mais ils devraient être mieux articulés les uns avec les autres, mieux expliqués, et surtout mieux évalués ! En tout état de cause, le fait d'augmenter en priorité les financements bilatéraux apparaît cohérent avec la volonté que nous exprimons tous de reprendre en main le pilotage politique de notre politique d'aide au développement. Une seconde manière d'y parvenir est d'améliorer l'évaluation. Le Président de la République a dit récemment : « Chaque euro doit être utilisé à bon escient. Aujourd'hui, l'évaluation reste marquée par son caractère lacunaire, par sa dispersion entre de multiples services- le principal appartenant à l'agence même dont il évalue les projets, à savoir l'AFD

ce qui ne fait qu'alimenter de constantes interrogations sur l'utilité de l'aide, son efficience et le devenir des projets dans le long terme. Dans ce domaine, sachons tirer parti de l'exemple de la commission indépendante pour l'impact de l'aide créée en 2011 par le gouvernement britannique ! Il faut notamment mettre davantage à contribution les cabinets d'expertise, fussent-ils privés, non pas, comme c'est le cas actuellement, pour qu'ils se livrent à une analyse polie et consensuelle sur tel ou tel programme, mais pour qu'ils produisent des évaluations indépendantes, incisives et sans concession. Enfin, monsieur le ministre, la décision de rapprocher Expertise France de l'Agence française de développement au sein d'un même groupe a été, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu précipitée au cours de l'été dernier. C'est vrai ! Au lieu de chercher à améliorer le modèle économique d'Expertise France, dont les résultats ont été remarquables, le Gouvernement a décidé de l'adosser à une AFD dont les moyens augmentent fortement. Cette solution de facilité pourrait engendrer d'autres problèmes, tant la culture de l'AFD est éloignée de celle d'une agence d'expertise technique. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous ce rapprochement, qui devra créer des synergies entre ces deux entités, mais aussi préserver l'autonomie d'Expertise France et sa capacité à poursuivre son action indispensable, notamment dans le domaine du continuum sécurité-développement ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, mes chers collègues, l'aide publique au développement est une composante essentielle de notre politique d'influence, mais également un impératif de justice et de solidarité internationale qui fait la fierté de la France. Néanmoins, force est de constater que nous avons échoué depuis quarante ans à remplir nos engagements internationaux en la matière. L'aide publique française n'a jamais dépassé 0,6 % du revenu national brut, contre un objectif fixé à 0,7 % par l'Assemblée générale des Nations unies en 1970. Elle est aujourd'hui plus proche de 0,4 %, ce qui semble insuffisant pour remplir les missions fixées au groupe AFD notamment, au Sahel et dans d'autres zones prioritaires. Face à ces défis, nous saluons l'initiative du Gouvernement, conformément aux orientations données par le Président de la République, de remettre la France sur la voie du respect de ses engagements. L'objectif intermédiaire de 0,55 % du RNB en 2022 nous semble réaliste, et l'augmentation de 4,7 % des crédits de la mission « Aide publique au développement » cette année, est un bon signal dans ce sens. Territoires regarde avec bienveillance cette évolution, mais restera vigilant quant au respect effectif de cet engagement. Dans un contexte budgétaire contraint, la tentation est en effet, souvent, de considérer l'aide au développement comme une variable d'ajustement. D'autres pays comme la Chine en ont au contraire fait une composante essentielle de leur diplomatie d'influence, en Afrique, et en Europe de l'Est notamment, avec un volontarisme politique fort et un effort financier important, appuyé sur de puissants opérateurs. Nous devons changer de logique dans notre approche de l'aide au développement. Elle est certes un impératif de solidarité, mais elle est aussi, et surtout, un investissement : un investissement dans l'avenir, un investissement dans la réussite, chez elle, d'une jeunesse qui s'abîme trop souvent dans une course folle vers l'Europe, un un investissement pour que la prospérité, demain, ne soit plus dans ces pays un rêve d'ailleurs, mais une réalité concrète. Avec cet objectif à l'esprit, il faut penser notre aide au développement d'une façon plus large, à la fois dans la définition des bailleurs, dans les types de projets financés et dans le pilotage des fonds. En ce qui concerne les acteurs, nous devons impérativement améliorer l'articulation entre l'État, les collectivités territoriales, les ONG et les entreprises ou fondations privées. L'avenir de l'aide publique au développement est aussi, peut-être, dans des partenariats entre les différents types de bailleurs, en fonction des expertises de chacun. En ce qui concerne les objectifs de l'aide au développement, nous voyons d'un bon oeil la convergence des processus « objectifs du développement durable et « financement du développement » sous l'égide des Nations unies. Ce rapprochement entre aide au développement et développement durable s'est matérialisé lors de la troisième conférence internationale sur le financement du développement à Addis-Abeba en juillet 2015. Le programme d'action d'Addis-Abeba adopté à son issue a envoyé un message fort sur l'importance du climat et de son intégration dans l'ensemble des politiques de développement. Les événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses ou les inondations sont des menaces importantes qui touchent l'ensemble des composantes- économique, sociale et politique Enfin, à propos du pilotage des fonds, deux divisions nous apparaissent structurantes et gagneraient à être éclaircies : tout d'abord, la division entre aides bilatérales et aides multilatérales- elles n'ont ni la même signification politique ni la même efficacité ensuite, la division des crédits entre deux programmes distincts, pilotés par deux ministères différents. Cet émiettement conduit à multiplier les instances de coordination. Il fait perdre à notre politique d'aide au développement à la fois lisibilité et efficacité. Sous réserve de ces quelques points de vigilance et en espérant, monsieur le ministre, que vous pourrez tenir compte de nos pistes de réflexion, le groupe Les Indépendants- République et Territoires votera ces crédits, qui poursuivent une remontée en puissance bienvenue de notre aide au développement.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

de Lyautey : quand je construis une école, je libère un bataillon. Aujourd'hui, c'est encore vrai : partout où nous menons des actions de développement, nous aidons à la lutte contre la radicalisation.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous abordons avec cette mission ce qui devrait être l'un des axes majeurs de la politique internationale de la France. notre pays n'a jamais été au rendez-vous de l'engagement international fixant à 0,7 % du PIB l'aide publique au développement. Longtemps, nous nous en sommes même éloignés. Pour la première fois, le budget inverse la trajectoire, et c'est tant mieux, mais en fixant d'emblée un objectif pour 2022 qui reste inférieur à 0,7 %.

Ce serait un signe fort de réorientation de notre politique extérieure, aujourd'hui clairement dominée par la militarisation de nos relations internationales. Si l'on ajoute la LPM, les OPEX et le niveau des ventes d'armes, dont nous sommes champions, on mesure à quel point l'APD fait figure de parent pauvre de notre politique internationale. Or c'est un grave contresens historique, tant le développement et la réduction des inégalités mondiales sont aujourd'hui les véritables clefs de la paix et de la sécurité collective mondiales. Je note toutefois que, adossées à l'effort budgétaire nouveau annoncé, la création d'un conseil de développement et la réactivation du conseil d'orientation stratégique de l'AFD constituent de premiers pas vers un nouveau pilotage de notre politique en la matière.

ce qui laisse planer un doute regrettable quant au respect de la trajectoire annoncée. Pour cette année, le Gouvernement annonce une progression de 1,4 milliard d'euros, mais la hausse réelle est plus limitée. En effet, 1 milliard d'euros crédité cette année ne pourra être décaissé que sur plusieurs années, et 270 millions d'euros proviennent d'une réécriture budgétaire, avec l'inscription dans la mission des fonds provenant initialement de la taxe sur les transactions financières. À ce propos, nous regrettons vivement la décision de diminuer la part de cette taxe dédiée à l'aide au développement. Elle laisse craindre de futures amputations du même type.

Ainsi, en réorientant la totalité du produit de la TTF et de la taxe sur les billets d'avion, et en lissant sur l'ensemble du quinquennat la hausse des crédits, nous aurions pu obtenir une trajectoire montant plus rapidement ; ce faisant, les objectifs finaux auraient

action est-elle bien à la hauteur de la situation ? Est-ce bien comprendre les enjeux du développement, quand la survie de la planète et le développement humain sont en cause ? Est-ce cette logique

Cette conception restrictive de l'APD est d'ailleurs contraire aux intentions premières de la déclaration de Paris et des principes de Busan. À nos yeux, la volonté exprimée d'inscrire dans l'APD des dépenses de sécurité et de défense

et inscrire ces investissements comme partie intégrante de l'APD. Si le secteur privé investit à l'étranger des fondations, c'est tant mieux. Mais l'État ne peut arguer de ces initiatives pour freiner les engagements propres du développement public.

la France et l'Europe sont aujourd'hui au coeur d'enjeux structurels majeurs : d'abord, la crise écologique ; ensuite, la pression des migrations économiques. Ces défis appellent, de par leur ampleur et leur pérennité, des réponses structurelles. Nous pouvons et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour adapter notre pays et trouver des solutions qui répondent aux effets de tels phénomènes. Mais nous devons aussi et surtout chercher à agir- je dis bien « agir -sur leurs causes, principalement dans les territoires où ils naissent. C'est en cela que l'aide au développement nous est essentielle. Il faut accompagner le développement des pays d'origine, pour permettre à leur jeunesse de demeurer sur place dans de bonnes conditions, de construire une famille et une vie décente. Nous éviterons ainsi que ces personnes viennent alimenter les flux de migration. De même, une réponse efficace à l'urgence climatique serait de proposer, à des pays qui polluent malgré eux énormément, des infrastructures urbaines, technologiques et énergétiques pourvues de technologies propres. L'enjeu est bien de limiter leur phase de dépendance aux énergies fossiles. À cet égard, faire du respect de l'accord de Paris un critère majeur dans la sélection des projets aidés par la France est une très bonne chose, et je tiens à saluer Ne l'oublions pas : cette politique ne doit pas seulement être justifiée par ce qu'elle pourrait nous rapporter, dans une logique purement comptable de retour sur investissement. Elle doit également résulter d'une responsabilité de solidarité à l'égard de nations dont les conditions de vie doivent être améliorées. nous saluons la progression significative des fonds alloués à l'aide publique au développement. Ils croissent en effet de 4,3 % en crédits de paiement et de près de 46 % en autorisations d'engagement, pour pas moins de 1,3 milliard d'euros supplémentaires. La montée en puissance de l'Agence française de développement démontre l'implication de notre pays dans le soutien au développement près de 40 milliards d'euros de bilan et environ 10 milliards d'euros d'engagements nouveaux en 2017, contre seulement 7 milliards d'euros en 2012. Je salue assurément cette progression. Essentielle à la politique d'influence de la France, l'aide publique au développement telle que mise en oeuvre par l'AFD doit en outre nous permettre de continuer à exister face au nouveau poids lourd qu'est la Chine ; ce grand pays est de plus en plus présent dans le monde, tout particulièrement en Afrique. Le Président de la République a annoncé que l'aide publique au développement passerait à 0,55 % du revenu national brut en 2022. en 2022. En conséquence, l'AFD devra encore accroître son activité, pour atteindre près de 18 milliards d'euros à cette échéance.

La volonté d'augmenter massivement les engagements ne doit pas aller à l'encontre de la pertinence des actions menées. Elle ne doit pas nuire à l'efficacité de l'aide. Nous devons ainsi veiller à ce que l'aide soit allouée à des projets oeuvrant effectivement au développement des régions concernées, en y associant pleinement les acteurs locaux. Les critères de sélection de ces projets doivent demeurer au coeur de notre stratégie d'aide. Nous y serons particulièrement vigilants. Enfin, j'aborderai la question de l'aide multilatérale au développement. admettre que nous en parlons peu, malgré son importance : nous versons beaucoup d'argent aux fonds multilatéraux, qui font sans doute du bon travail, mais dans une opacité que je qualifierai de regrettable.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour 2019, le budget de l'APD connaît une hausse substantielle, et je m'en félicite. Mais n'est-ce pas là une augmentation en trompe-l'oeil ? Le chiffre de 1 milliard d'euros d'augmentation est impressionnant, mais il s'agit d'autorisations d'engagement. En crédits de paiement, cette hausse se limite à 130 millions d'euros. Cela masque un recul grave. La taxe sur les transactions financières, jusqu'alors affectée à 50 % à l'APD, ne le sera plus qu'à hauteur de 32 %. Si cette déviation du flux de la TTF est, cette année, compensée budgétairement, donnant la possibilité de communiquer sur une augmentation de budget largement rien ne dit que tel sera le cas dans le futur. Le risque est d'entériner le principe d'une baisse de l'affectation de ce financement innovant. Pour aller plus loin dans la recherche de financements innovants, pourquoi ne pas, par par exemple, taxer les cargos, qui acheminent plus de 90 % des marchandises de la planète et dégagent une pollution massive ? Il y a un certain manque de réalisme dans la réaffirmation de la cible de 0,55 % du RNB en fin de quinquennat, objectif déjà peu ambitieux par rapport à nos engagements anciens de 0,7 %, auxquels nombre de nos partenaires européens sont déjà parvenus. Il risque fort de ne pas être tenu, car la trajectoire proposée fait reposer l'essentiel de l'effort sur la fin du quinquennat. Nous étions à 0,43 % en 2017, nous ne serons qu'à 0,44 % en 2019, en 2019, loin de l'objectif affiché. Je salue en revanche le début de rééquilibrage entre dons et prêts. Octroyer des prêts n'est pas la raison d'être de notre APD, surtout quand il s'agit de pays ayant les moyens de financer leur propre développement, voire d'investir dans les pays du Sud, comme la Chine, encore fortement bénéficiaire de notre APD, qui investit massivement en Afrique sans se préoccuper de normes sociales ou environnementales. Les aides sous forme de dons, privilégiées par les agences de développement britanniques et allemandes, favorisent des projets en faveur de biens communs comme l'environnement, la santé ou l'éducation. Cela fait des années que je plaide pour un renforcement du soutien français à l'éducation, notamment celle des filles, et je ne peux que me réjouir qu'il soit enfin élevé au rang de priorité. Les bienfaits des investissements dans l'éducation sont en effet nombreux, tant en matière de développement économique que d'égalité femmes-hommes, de santé, de lutte contre le changement climatique ou de limitation de la pression migratoire. Mais l'APD délivrée sous forme de dons est aussi plus coûteuse pour le contribuable, d'où une exigence accrue en matière de contrôle et de recevabilité, surtout au regard des contraintes budgétaires qui pèsent sur l'ensemble des autres budgets de l'État. Pour renforcer le contrôle et l'évaluation, nous avons besoin de définir avec beaucoup plus de rigueur des indicateurs assortis de cibles chiffrées. C'est notamment indispensable pour évaluer notre impact sur des enjeux transversaux tels que l'égalité de genre ou la cohérence de nos actions en matière d'empreinte carbone. Autre enjeu sur lequel notre budget manque de vision à long terme : la francophonie. La France ne consacre que 32 % de son APD à des pays francophones- presque deux fois moins que ce que le Royaume-Uni

Une plus grande implication dans l'aire francophone serait doublement vertueuse, puisqu'elle permettrait de renforcer notre ancrage dans une zone en forte croissance tout en nourrissant cette dernière. Dans un contexte de forte concurrence internationale, notamment chinoise, il est important de jouer toutes nos cartes. Je défendrai tout à l'heure un amendement visant à sécuriser des financements pour notre audiovisuel extérieur. J'estime également qu'un déploiement financier de l'AFD réalisé sur fond d'étranglement budgétaire du Quai d'Orsay est contre-productif. Si nous voulons sortir du saupoudrage et du court-termisme, nous devons intégrer notre aide au développement dans un dialogue diplomatique de qualité. À cet égard, le financement de 50 millions d'euros au gouvernement gambien, n'est pas le meilleur exemple de démocratie, apparaîtrait presque comme une provocation au regard des coupes budgétaires drastiques imposées à notre ministère des affaires étrangères collègue ! Je conclurai simplement en rappelant combien nous devons être vertueux et combien notre aide au développement devrait aussi servir d'élément déterminant dans notre action diplomatique extérieure, avec un contrôle accru.

Or, pas plus que le budget pour 2018, le budget pour 2019 n'engage la France sur une trajectoire crédible vers cet objectif. Certes, cette trajectoire prévoit une forte augmentation en fin de quinquennat, mais on peut s'interroger sur cette accélération très forte à partir de 2020 quand on sait que l'APD a souvent servi, par le passé, et sous tous les gouvernements, de variable d'ajustement en cas de difficultés budgétaires. nous sommes loin d'allouer à l'APD 0,7 % du revenu national brut ; 0,7 %, ce chiffre qui fait consensus dans les instances internationales et que d'autres pays européens ont déjà atteint : la Norvège, le Royaume-Uni, le Danemark ou encore l'Allemagne.

faiblesse des dons conduit depuis longtemps l'APD française vers les pays les plus solvables ; les pays les plus pauvres ne bénéficient, eux, que d'un quart de l'aide française, les autres étant notamment des pays émergents, comme la Chine, le Brésil ou encore l'Afrique du Sud.

Les deux tiers de la hausse des autorisations d'engagement de l'APD d'ici à 2022 devront contribuer à la composante bilatérale de l'aide au développement. Parallèlement, les dons progresseront aussi, l'AFD devant bénéficier dès 2019 de plus de 1 milliard d'euros d'autorisations d'engagement.

d'euros et les autorisations d'engagement, en forte hausse, ne seront mises en oeuvre que sur plusieurs années. L'aide réelle aux pays les plus pauvres, notamment ceux du Sahel, dépendra donc du renouvellement de ce niveau élevé d'autorisations d'engagement au cours des prochaines années.

concerne les prêts, le plan de croissance rapide des engagements de l'AFD pose deux questions. Premièrement, la majorité de ces engagements correspond à des prêts à taux de marché ou faiblement bonifiés, contractés avec des pays à revenu intermédiaire ou des pays émergents. Je pense à la Turquie, au Maroc, à la Colombie, à l'Inde, au Brésil, à l'Égypte, ou encore à la Jordanie. Or, dès 2018, la forte dégradation des capacités d'emprunt de plusieurs de ces États risque de rendre l'objectif de croissance des engagements de l'AFD plus difficile à atteindre. Deuxièmement, si l'AFD parvient à augmenter encore ses prêts, ne risque-t-on pas d'observer une diminution de la qualité de ces engagements, avec des projets qui ne répondraient pas forcément à toutes les exigences environnementales, sociales ou de bonne gouvernance, de démocratie, que l'AFD doit respecter ? Dans le même ordre d'idées, ce plan de croissance va obliger l'Agence à demander l'extension de son mandat à de nouveaux pays, au risque de nuire à la cohérence de la politique d'aide au développement.

au développement qu'à hauteur de 30 %. Jusqu'à présent, la TTF était allouée pour 528 millions d'euros au Fonds de solidarité pour le développement, le FSD, et pour 270 millions d'euros à l'AFD. Or le projet de loi de finances pour 2019 supprime la part affectée à l'AFD. Marie-Françoise Perol-Dumont en a parlé à l'instant.

par des moissons de chiffres et de comparaisons traduisant notre approbation, nos craintes ou nos réserves. Permettez-moi de déroger à cette tradition en abordant les crédits consacrés à l'aide publique au développement. Les montants de ces crédits sont peu de choses au regard des grands postes de dépenses de l'État, mais ils ont, à mes yeux, une importance déterminante sur le sens de la politique mise en oeuvre par notre pays. Comme la plupart d'entre nous, je me félicite que cette politique publique bénéficie d'une hausse d'environ 4,7 %, les crédits de paiement augmentant de 127 millions d'euros et les autorisations d'engagement, Je me remémore le discours du Président de la République prononcé à Ouagadougou en novembre 2017. Je me souviens plus précisément d'une phrase : « J'ai pris l'engagement d'avoir une France au rendez-vous du défi de

car cette hausse de crédits est loin d'être négligeable au regard du contexte économique auquel notre pays est confronté. Elle est d'autant plus significative qu'au niveau mondial l'aide publique au développement, d'un montant de 146 milliards de dollars, est en baisse de 0,6 %. À l'heure où les crises liées au changement climatique s'ajoutent aux guerres et conflits, nous pouvons être fiers de joindre actes et paroles, même si bien des efforts restent à accomplir. Je n'insisterai pas non plus sur les équilibres entre autorisations d'engagement et crédits de paiement structurant les moyens alloués à cette politique publique. Ils s'expliquent par l'augmentation de notre contribution au Fonds européen de développement et trouvent aussi leur justification dans les fluctuations des autorisations d'engagement auxquelles nous avons à nous adapter. Ayant fermement critiqué l'an passé, à cette même tribune, le risque de déclassement de notre pays, comment ne pas être réconforté en constatant l'inversion de la trajectoire inscrite dans le nous laisse entrevoir la possibilité d'atteindre le chiffre de 0,55 % de notre revenu national brut consacré à cette politique en 2022 Les esprits chagrins feront remarquer que nous sommes loin des objectifs électoraux du Président de la République. Pour ma part, je préfère voir le verre à moitié plein d'un chapitre budgétaire qui inverse « à la hausse » la courbe du montant de nos aides, alors que l'Allemagne ou le Royaume-Uni ont déjà atteint ce seuil de financement. Si je salue notre trajectoire, en refusant de m'adonner à la litanie des indices et des chiffres, c'est pour insister sur le sens que nous devons donner à cette politique. Nous avons tous entendu

la réalité infirme ces jugements, et les besoins pour lutter contre la faim, la pauvreté, permettre à l'accès à l'eau et favoriser l'éducation rendent cette aide indispensable. Même imparfaite, même insuffisante, elle est l'une des pièces essentielles au travers de laquelle nous traduisons un devoir de solidarité. À l'heure où la France traverse une grave crise et où nos concitoyens nous demandent de penser à leur pouvoir d'achat, renforcer l'aide publique au développement, c'est dire clairement que rien ne pourra se faire ici si l'on ne prend pas soin de ceux et celles qui souffrent aussi ailleurs. N'oublions pas, mes chers collègues, les 17 000 enfants qui meurent chaque jour dans le monde Plus que jamais, le développement constitue un enjeu géopolitique fort. Monsieur le ministre, malgré les réserves que je viens de formuler, parce que ces crédits sont orientés à la hausse et parce que l'aide publique au développement n'est qu'une part du soutien que la France apporte aux pays les plus fragiles, le groupe du RDSE votera ce budget. La

sur une mission qui, chacun a bien voulu le reconnaître, enregistre une progression très significative de ses crédits. Le programme 209

a décidé, pour financer les annonces récentes du Premier ministre, un ajustement à la baisse de certains plafonds budgétaires. Or, pour ce qui concerne mon ministère, nous avons appris à la fin du mois de novembre que la contribution française au FED serait inférieure à la prévision initiale, ce qui nous permet de porter l'ensemble de l'ajustement qui nous est demandé sur le programme 209, sans qu'aucune des actions prévues soit remise en cause,

des actions pour résorber les fragilités en zone de crise, la lutte contre le changement climatique et l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle permettra aussi d'affirmer nos choix géographiques

j'ai fait, vous le savez, une priorité. Comme je m'y étais engagé l'an dernier, les crédits de gestion et de sortie de crise augmentent, cette année encore, de 14 millions d'euros, pour atteindre 100 millions d'euros. À ce titre, le Fonds d'urgence humanitaire sera porté à 45 millions d'euros et notre aide alimentaire programmée sera également renforcée. Nous devenons enfin un acteur humanitaire significatif et sortons d'une situation où nous investissions dans ce secteur moins qu'un pays comme la Belgique- j'avais eu l'occasion de vous le dire l'année dernière. Je souhaite que le débat

soit l'occasion de réfléchir aux moyens permettant de suivre l'utilisation de ces ressources importantes. Il convient en effet de disposer de moyens de pilotage et d'évaluation adaptés à l'effort consenti.

Premièrement, l'AFD sera en première ligne dans la mise en oeuvre de ces moyens nouveaux. Nous renégocierons en 2019 sa rémunération. Les ressources ainsi dégagées abonderont le Fonds de solidarité pour les partenariats innovants, le FSPI, qui est facile d'usage, très facile d'usage, très réactif et généralement à la main des ambassadeurs pour financer des programmes de volume modeste ou dans leur phase initiale. C'est ainsi que ce fonds a permis les premiers travaux de conception du futur campus franco-sénégalais de Dakar. Deuxièmement, les nouveaux financiers accordés à l'AFD doivent conduire à renforcer son pilotage. Dans la réflexion que nous menons pour élaborer le projet de loi, plusieurs propositions formulées par le député Hervé Berville dans le rapport qu'il nous a remis ont retenu notre attention. Comme il l'a proposé, nous envisageons de créer un conseil de développement sous l'autorité du Président de la République. Par ailleurs, il sera bien précisé dans le projet de loi qu'il reviendra au ministre chargé de la coopération,

a demandé au Président de la République, lors de la réunion du G 20 à Buenos Aires, que la France joue un rôle majeur dans le cadre du sommet sur le climat de septembre 2019 qu'il organisera à New York. Nous aurons la responsabilité, avec la Jamaïque, d'identifier les enjeux de financement du futur et de faire en sorte que les outils de financement soient au

de loi de finances à l'Assemblée nationale, nos collègues députés ont augmenté plusieurs dépenses, notamment les crédits relatifs à la prime pour l'emploi. Au total, 236 millions d'euros ont dû être financés en seconde délibération par la « solidarité gouvernementale

de 6,7 millions d'euros. Un second amendement, qui a déjà été déposé, vise à majorer du même montant les crédits de la mission « Action extérieure de l'État ». Ce choix vient du fait que les appels de la Commission européenne pour le Fonds européen de développement devraient être moins importants que prévu,

monsieur le ministre, quel est le montant exact de cette économie de constatation ? Permettra-t-elle également d'absorber la « première minoration » du programme 209 ?

ainsi libellé : La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Cet amendement vise à permettre, par la création d'une ligne de crédits dans le programme 209, « Solidarité à l'égard des pays en développement », le financement des actions d'aide publique au développement réalisées par France Médias Monde. Cet opérateur de l'action audiovisuelle extérieure de la France diffuse sur ses antennes linéaires- RFI, France 24, MCD -et numériques des programmes de service public destinés aux populations des pays en développement les plus pauvres, notamment en Afrique et dans les zones de crise. Nombre de ces programmes portent ou sont susceptibles de porter sur des domaines considérés comme prioritaires par le CICID, le comité interministériel de la coopération internationale et du développement : éducation, apprentissage du français, santé, environnement ... Il s'agit de reconnaître cette mission de service public. Nombre de médias internationaux, desquels figure la BBC World Service, bénéficient, à ce titre, de financements budgétaires de leur gouvernement. Afin d'assurer la pérennité de ce financement, il est proposé de doter cette ligne d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement. Les montants, 12 millions d'euros en autorisations d'engagement et 4 millions d'euros en crédits de paiement, correspondent au besoin de financement nécessaire, voire indispensable, pour maintenir la production et la diffusion de ces programmes en Afrique, notamment dans les langues locales, et de développer de nouvelles émissions thématiques de service public. Cette action est financée par une réduction d'un même montant sur les crédits du programme 110, « Aide économique et financière au développement ». Il s'agit vraiment, monsieur le ministre, d'une priorité au regard d'un environnement extrêmement compétitif, au sein duquel nous avons vraiment besoin de nous affirmer. Sinon, nous risquons de perdre énormément de parts de marché que nous aurons beaucoup de mal à récupérer par la suite.

ont diminué en 2018 et connaissent une nouvelle baisse en 2019 de 2 millions d'euros. En conséquence, le présent amendement vise à accorder 12 millions d'euros supplémentaires à l'audiovisuel extérieur français.

Certes, CFI est une filiale de FMM, mais il n'y a pas de fongibilité des budgets. Ainsi, ces crédits permettraient non pas de maintenir la production et la diffusion de programmes en Afrique, contrairement à ce qu'indique l'objet de cet amendement, mais de financer des missions de coopération technique dans les pays en développement. Les missions de CFI consistent notamment à promouvoir la diffusion par les médias locaux de contenus sur les enjeux du développement durable et à soutenir les instances locales de régulation et l'optimisation des grilles des programmations des chaînes de ces pays. Je précise que la dotation

Jean-Pierre Leleux souhaite également les majorer de 3 millions d'euros. Je comprends la préoccupation de nos collègues pour l'audiovisuel public. Toutefois, il est important de maintenir une certaine lisibilité : l'aide publique au développement est, au sens de l'OCDE, un agrégat complexe. N'ajoutons pas de la complexité en demandant à l'aide publique au développement de financer l'audiovisuel, sinon, demain, on demandera aussi à cette mission de financer les universités, la vie étudiante, l'accueil des réfugiés, la recherche agricole, la diplomatie culturelle, la gendarmerie et même certaines des bases militaires. Ma chère collègue, je vous invite à

de récupérer un peu plus de 80 millions d'euros. Malheureusement, je le dis tout de suite à notre collègue Assouline, l'Assemblée nationale n'en veut pas, et le Gouvernement non plus. Il le fera donc supprimer

Je considérais que la baisse du budget de l'audiovisuel public d'environ 80 millions

de la suite du débat sur le projet de loi de finances, grâce à l'amendement que j'ai présenté, il y a l'argent suffisant pour habiller France Médias Monde sans déshabiller ni l'AFD ni le reste du service public de l'audiovisuel.

a urgence : le budget de France Médias Monde est en retrait de 7 millions d'euros par rapport aux engagements pris par le Gouvernement dans le contrat d'objectifs et de moyens. C'est énorme ! Cette situation d'urgence fait que, si France Médias Monde n'obtient pas au début de 2019 des crédits suffisants, elle se trouvera rapidement dans l'obligation de supprimer un certain nombre d'émissions, à un moment où jamais il n'a été aussi important d'avoir une présence médiatique

Doté d'un peu moins de 3 milliards d'euros en crédits de paiement, ce budget est relativement sobre compte tenu des missions qu'il doit remplir. L'exercice 2019 se caractérise par la poursuite des efforts budgétaires réalisés ces dernières années par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit 2,9 milliards d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. À périmètre courant, les crédits de la mission diminuent ainsi de 4,3 %.

Cette baisse est moins importante que prévu par la loi de programmation des finances publiques votée au mois de juillet. De ce point de vue, la distinction entre périmètre courant et périmètre constant est utile au Gouvernement, car le périmètre courant permet d'afficher un respect du plafond fixé par la loi de programmation des finances publiques à 2,75 milliards d'euros, hors contribution au compte d'affectation spéciale « Pensions

Mon examen a porté plus précisément sur le programme 105 de la mission, sur lequel reposent les dépenses de personnel et de fonctionnement des réseaux diplomatique et consulaire ainsi que les contributions internationales. J'ai aussi examiné les crédits relatifs à l'organisation du G7 par la France en 2019. Le programme 105 est au coeur de la reconfiguration des réseaux de l'État à l'étranger souhaitée par le Président de la République. En effet, à partir de 2019, le programme 105 devient le programme support de l'ensemble des opérateurs et ministères à l'étranger. Par conséquent, il devient affectataire de l'ensemble des immeubles possédés par l'État à l'étranger, ce qui devrait contribuer à l'élaboration d'une stratégie interministérielle plus efficace de gestion du parc immobilier de l'État.

Ce nouvel exercice d'effort budgétaire pour nos postes à l'étranger est bienvenu. Le cloisonnement des fonctions supports ne permet pas d'établir une vision transversale des moyens mis en oeuvre. Je regrette toutefois que la conduite de la réforme ait éclipsé une réflexion sur la valeur ajoutée de certains postes diplomatiques et consulaires, au nom du choix de l'universalité du réseau. Je souhaiterais appeler votre attention sur plusieurs points de vigilance. Premièrement, l'érosion des moyens humains du ministère n'empêche pas le dynamisme des dépenses de personnel. Depuis dix ans, le nombre d'équivalents temps plein travaillé a diminué de près de 12 %, mais les dépenses de personnel ont augmenté de 23 %. Une réflexion sur la gestion des ressources humaines du ministère doit impérativement être enclenchée. Les documents budgétaires montrent par ailleurs un dérapage des dépenses de personnel pour l'exercice 2018, ce qui expliquerait l'écart avec la trajectoire définie par la loi de programmation des finances publiques. Comment expliquez-vous que les dépenses de personnel, en 2018, soient près de 30 millions d'euros supérieures aux prévisions ? les contributions internationales et européennes devraient diminuer de 70 millions d'euros environ entre 2018 et 2019, sous l'effet de l'évolution des opérations de maintien de la paix.

la politique immobilière du ministère doit faire l'objet d'un pilotage renforcé. À la fin de 2016, son parc immobilier était estimé à 4,3 milliards d'euros. L'immobilier du ministère va être mis à contribution pour financer les dépenses de sécurisation des implantations à l'étranger. Les avances du compte d'affectation spéciale « Gestion immobilière de l'État » devraient représenter 100 millions d'euros, qui devront être remboursés par les produits de cession. Or ceux-ci ne cessent de se réduire et ne devraient représenter que 30 millions d'euros en 2018. Comment comptez-vous rembourser ces avances et à quelle échéance ? Enfin, concernant le programme 347, « Présidence française du G7 », le coût estimé s'élève à 36,4 millions d'euros, 3,2 millions d'euros au titre des dépenses de protocole. Ce coût est supérieur à celui de l'organisation du G20 en 2008, à Deauville, même en tenant compte de l'inflation. Par conséquent, je présenterai deux amendements visant respectivement à aligner le coût du G7 sur celui du G20 de 2008 et à réduire les dépenses liées à l'organisation de la réunion des ministres des affaires étrangères du G7, qui ne figurent pas dans ce programme et sont rattachées aux dépenses protocolaires. Le projet de budget pour 2019 de la mission « Action extérieure de l'État » a été critiqué en raison des réformes structurelles qui ont été annoncées, notamment de 10 % de la masse salariale d'ici à 2022, qui inquiète beaucoup. Il me semble qu'un examen attentif permet plutôt de souligner une relative préservation de nos moyens à l'étranger pour 2019 et de mettre en évidence l'existence de certaines marges de manoeuvre budgétaires, sous réserve des points de vigilance dont je vous ai fait part.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à la suite de Vincent Delahaye, je vais brièvement vous présenter les programmes de la mission « Action extérieure de l'État » qui concernent,

Cependant, la réduction des emplois du ministère de l'Europe et des affaires étrangères reste préoccupante. La répartition des crédits ne semble donc pas totalement en accord avec la volonté d'avoir de grandes ambitions diplomatiques et une vocation universelle

Autre marqueur de modernisation : la mise en place du vote électronique sera effective dès le prochain scrutin européen. Le budget alloué à l'organisation des élections européennes est de 3,5 millions d'euros, soit une somme équivalente à celle de 2014. Cela ne devrait donc pas poser de difficultés.

Il est intéressant de noter que près de la moitié des subventions sollicitées sont destinées à soutenir un projet éducatif. Nous pourrons certainement mieux en juger l'an prochain- nous pourrons tirer le bilan de l'année 2018 -, en espérant que les crédits pour 2019 pourront être intégralement consommés, car la campagne d'examen d'examen des demandes de subventions commencera plus tôt. Mais nous pouvons d'ores et déjà constater que ce dispositif de remplacement de la réserve parlementaire semble fonctionner Concernant les acteurs culturels et l'enseignement ainsi que les opérateurs chargés de la politique d'influence de notre pays, la stabilité des crédits apparaît davantage comme un sursis bienvenu, qui n'enlève rien à la nécessité d'établir une stratégie claire de développement du français pour les années à venir. À la suite des annonces du Président de la République sur le plan Langue française, en mars dernier, l'Institut français bénéficiera de 2 millions d'euros supplémentaires. Il faut saluer cet effort, en ajoutant que des précisions doivent encore être apportées, notamment, sur le rapprochement entre l'Institut français et la Fondation Alliance française, qui a été acté lors de l'examen du projet de loi de finances pour Les subventions et les emplois des autres opérateurs sont, eux, maintenus à un niveau équivalent à celui de 2018, ce qui marque la volonté de préserver leurs missions en matière d'attractivité de notre pays.

Il s'agit d'un des plus grands réseaux d'enseignement public à l'étranger au monde, ce qui en fait un atout très précieux pour la scolarisation des enfants français à l'étranger et pour le rayonnement de notre pays. Si la préservation, cette année, du budget de l'enseignement français à l'étranger semble positive, elle ne saurait occulter d'importantes tensions. L'annulation d'une partie de la subvention de l'AEFE, à hauteur de 33 millions d'euros, à l'été 2017, avait mis en évidence la difficile équation budgétaire de l'Agence. Celle-ci fait face, depuis de nombreuses années, à une hausse structurelle de ses dépenses parallèle à un désengagement progressif de l'État. Dans ces conditions, les familles sont de plus en plus mises à contribution et les frais de scolarité par élève ont beaucoup augmenté ces dernières années. La stabilité budgétaire, pour 2019, était donc indispensable. Il faut saluer sa concrétisation. Pour faire face aux difficultés, en effet, l'AEFE a réduit le nombre de postes d'enseignants et d'encadrement qu'elle finance : elle a supprimé 80 postes d'expatriés et 100 postes d'enseignants résidents cette année ; elle prévoit d'en supprimer 166 autres en 2019.

Elles sont en outre contradictoires, en apparence en tout cas, avec l'objectif de doublement du nombre d'élèves scolarisés dans le réseau d'ici à 2030.

Pour conclure, je dirai que ce budget, s'il est tout à fait convenable du point de vue de l'examen de cet exercice budgétaire, semble insuffisant à long terme au regard des ambitions exprimées.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 2019, les efforts en faveur de la sécurité extérieure au sens large se poursuivent.

qui constitue notre « premier bouclier au loin », illustration parfaite du entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. Il s'agit là d'un rééquilibrage, à un étiage encore bas, mais essentiel à la cohérence de notre politique. Après une forte baisse, les crédits retrouvent le niveau qu'ils avaient voilà dix ans, soit 104 millions d'euros. Nous avons dans ce domaine deux recommandations. La première consiste à veiller à ne pas imposer une réduction d'effectifs : il faut laisser la direction gérer une baisse de la masse salariale et retrouver ainsi une certaine souplesse au lieu de prévoir la suppression de vingt équivalents temps plein de 2019 à 2022. La deuxième concerne la loi d'orientation et de programmation de l'aide publique au développement, qui doit permettre d'assurer le financement du entre la sécurité et le développement, en finançant, si possible, hors programme 105 les actions de la DCDS renforçant les capacités des États partenaires dans les domaines de la sécurité intérieure et de la protection civile. protection civile. En 2019, les crédits budgétaires dédiés à la sécurisation des emprises françaises à l'étranger diminuent, passant de 75 millions à 44 millions d'euros. Cette réduction de crédits est compensée par une avance de 100 millions d'euros sur deux ans du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Pour 2019, les crédits du programme 151 enregistrent une modeste augmentation, de 1,5 %, qui ne doit pas dissimuler le régime d'austérité imposé à notre réseau consulaire. De fait, cette hausse s'explique avant tout par une réévaluation des crédits de titre 2, réévaluation destinée à compenser leur sous-évaluation l'année dernière. Il ne s'agit en aucun cas d'augmenter les effectifs, puisque le programme 151 perdra trente-sept équivalents temps plein en 2019, afin de se afin de se conformer aux objectifs du projet Action publique 2022 de réduction des réseaux de l'État à l'étranger. Hors titre 2, les Hors titre 2, les crédits du programme diminuent de 2,6 %, malgré des transferts de crédits à son profit liés à la nécessité de préparer les élections européennes de mai 2019, à l'abondement du dispositif STAFE, créé pour compenser la suppression de la réserve parlementaire, et, dans une moindre mesure, au rapatriement de crédits d'adoption en provenance du programme 185. C'est ainsi que certaines lignes subissent des ajustements. C'est le cas de l'aide sociale distribuée par les comités consulaires, en diminution de 1,9 million d'euros. Cette diminution, nous dit-on, s'expliquerait par une baisse du nombre d'allocataires. Nous en doutons un peu. Je rappelle que ces aides, souvent d'un faible montant, n'en sont pas moins importantes pour nos compatriotes à l'étranger en difficulté. Ce sont donc les plus modestes qui risquent de souffrir. De même, la dotation destinée aux bourses scolaires, qui était stable l'an passé, se trouve diminuée de 5 millions d'euros, à 105,3 millions d'euros, au motif qu'il sera possible de puiser dans la soulte de l'AEFE pour compléter si besoin. Certes, cette soulte constitue une réserve confortable qui a de surcroît l'avantage de se reconstituer grâce aux effets de change, mais cela pourrait ne pas durer. Qu'adviendra-t-il si les circonstances sont moins favorables ? La baisse de l'enveloppe budgétaire sera-t-elle réversible ? Ma crainte est que ne se produise un « effet de cliquet ». Les suppressions d'emplois prévues en 2019- elles ne sont que la première marche effort appelé à s'accentuer les années suivantes -ne seront possibles qu'au prix de nouvelles mesures de rationalisation : regroupement d'activités, par exemple en matière de transcription de l'état civil, ajustement au strict minimum des effectifs des « postes à gestion simplifiée », poursuite de l'externalisation du traitement des demandes de visas, transformation de postes d'agents titulaires en postes d'agents de droit local ... Je le souligne, cette manoeuvre n'est pas sans risque dans certains pays. Par ailleurs, l'administration consulaire continuera à moderniser à dégager des gains de productivité, à travers des projets tels que le paiement en ligne des droits de chancellerie, la pré-demande en ligne des passeports ou encore le lancement d'une expérimentation visant à permettre la transmission dématérialisée des actes d'état civil aux Français de l'étranger.

part de mon inquiétude quant à la réduction continue des moyens d'une administration efficace et appréciée, qui- nous avons déjà eu l'occasion de le dire -ne pourra pas indéfiniment faire plus avec moins. Au final, c'est la capacité d'influence et de rayonnement de la France dans le monde qui en sera amoindrie.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de mettre l'accent sur quatre points importants, je souhaite je souhaite rappeler toute l'importance du programme 151, qui représente les services publics aux Français de l'étranger. Le premier point concerne le dispositif de soutien au tissu associatif des Français de l'étranger, dit STAFE. Bien que faisant suite à la suppression de la réserve parlementaire, celui-ci accuse une baisse d'un tiers des crédits consacrés, passant de 3 millions à 2 millions d'euros. Par ailleurs, nous regrettons qu'aucune place n'ait été prévue pour les parlementaires dans ce dispositif, contrairement au précédent. Très bien Pour autant, le bilan de la première campagne semble encourageant. Monsieur le ministre, quels enseignements en tirez-vous ? Quelles adaptations envisagez-vous pour la suite ? Le deuxième point, également abordé par mon corapporteur Jean-Pierre Grand, est celui des bourses scolaires et des aides aux familles.

pour les citoyens européens présents sur le territoire britannique au terme de la période de transition fixée au 31 décembre 2020. Ils pourront continuer à vivre, travailler ou étudier dans les mêmes conditions qu'actuellement. Je veux néanmoins me faire l'écho des préoccupations exprimées par un certain nombre d'associations de ressortissants européens résidant au Royaume-Uni. Elles s'inquiètent de la capacité de l'administration britannique à procéder, sans erreur

réflexions multiples, encore inabouties. Un rapprochement de l'Institut français et de la Fondation Alliance française est en cours. L'enseignement français à l'étranger doit être développé. Le Président de la République a présenté un plan ambitieux pour la langue française et le plurilinguisme. Dont acte Mais les moyens sont-ils au rendez-vous ? Je concentrerai mes remarques sur l'AEFE. La subvention est stable, après une année difficile. Plusieurs mesures très contraignantes pour les établissements Je vous rappelle l'augmentation du taux de la participation française complémentaire sur les frais de scolarité, à 9 %. On nous dit que ce sera 7,5 %.

Lorsque l'État se désengage, ce sont donc automatiquement les familles qui paient. Or elles paient de plus en plus, et de plus en plus de familles françaises à l'étranger à revenus modestes ont des difficultés.

des écoles françaises de l'étranger, l'ANEFE, ait stoppé ses activités de prêts garantis par l'État aux établissements ? Tout semble concourir à compliquer la tâche des établissements français à l'étranger,

Au moment où se dessine un mouvement de restitution aux pays africains de biens mal acquis sur l'initiative du Président de la République, au moment de l'amorce d'un processus d'inventaire de la colonisation, notamment de la colonisation de l'Algérie, cette hausse brutale du montant d'inscription constitue un très mauvais signal. En renonçant à accueillir une majorité d'étudiants africains, la France renonce à toute relation privilégiée avec les cadres africains de demain. ces futurs cadres sont convoités par de nouveaux acteurs, comme la Chine, l'Inde et la Russie. En 2018, les étudiants africains inscrits en Chine devraient atteindre le chiffre de 80 000. Ils y bénéficient de la scolarisation et du logement gratuits ainsi que de bourses de 400 euros mensuels. Si l'Europe et la France restent leur priorité, nous perdons du terrain, notamment au profit de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis ou de la Turquie, qui proposent des bourses dans des universités islamiques.

un renoncement. On abandonne à d'autres pays le soin de former les cadres de demain. Ce renoncement va aggraver la perte d'influence de la France sur le continent africain, la déception, le dépit et, demain, le rejet de notre pays par la jeunesse du continent le plus jeune du monde.

doivent vous alerter, monsieur le ministre. Il faut absolument revoir cette décision funeste pour le rayonnement culturel et économique de la France, mais aussi pour la francophonie.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les crédits destinés à notre diplomatie culturelle et d'influence ont été les grands sacrifiés du quinquennat de François Hollande de plus de 750 millions d'euros en 2012, ils sont tombés à moins de 685 millions d'euros cinq ans plus tard, soit une baisse inédite de près En cette deuxième année du quinquennat d'Emmanuel Macron, nous voyons déjà ce que sera la marque de fabrique du nouveau Président de la République : de grandes envolées, de beaux discours, des intentions louables, trente-trois mesures dans le plan Langue française et plurilinguisme ... Qui d'entre nous ne serait pas derrière le Président de la République pour « donner un nouvel élan à notre diplomatie culturelle », comme il s'y est engagé ? Personne Mais, derrière les beaux discours, derrière les grandes envolées lyriques, quand on regarde dans le détail le budget, qui est le reflet de la véritable politique menée par le Gouvernement, que voit-on ? Des crédits durablement maintenus au niveau bas atteint en 2017, comme une confirmation, une acceptation, de la politique menée durant le précédent quinquennat ! Et les années à venir risquent d'être particulièrement douloureuses, le Gouvernement ayant annoncé dans le cadre du plan Action publique 2022 la réduction de 10 % de la masse salariale de l'ensemble des réseaux de l'État à l'étranger d'ici à 2022 Dans ces conditions, si l'on regarde les opérateurs de notre diplomatie culturelle, comment mettre en oeuvre dix-sept des trente-trois mesures du plan Langue française et plurilinguisme avec seulement 2 millions d'euros supplémentaires non reconductibles et aucun emploi pour l'Institut français ? Comment doubler le nombre d'étudiants internationaux accueillis en France avec un budget inchangé pour Campus France ? Surtout, comment doubler le nombre d'élèves scolarisés dans notre réseau à l'étranger, avec un budget également inchangé pour l'AEFE ? Atteindre les 700 000 élèves dans le réseau en 2030, comme l'a annoncé le Président de la République, c'est l'équivalent de l'ouverture de quarante-huit établissements tous les ans pendant treize ans. Est-ce un objectif vraiment raisonnable ? Je m'interroge aussi sur le devenir de la Fondation Alliance française, qui, si elle a échappé à la disparition, est néanmoins profondément dévitalisée dans l'opération de rapprochement avec l'Institut français.

Mais pour combien de temps encore, au regard des coupes budgétaires drastiques dont fait l'objet notre réseau à l'étranger ? Mes chers collègues, vous le voyez, ma frustration est grande et mes réserves sont immenses. La commission de la culture, sans enthousiasme aucun, mais au vu de la stabilité de ce programme, a néanmoins choisi d'émettre un avis favorable à l'adoption

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quoi de plus essentiel en vérité, malgré leur modestie, que les crédits du Quai d'Orsay ? Ce budget porte en effet l'action diplomatique de la France dans le monde. Or la voix de la France est aujourd'hui absolument primordiale. Le monde est confronté à une forme de « chaos » géopolitique. il y a l'aggravation des menaces. Menaces de la force, on le voit ces jours-ci en mer d'Azov, comme hier en Crimée, mais aussi en mer de Chine, dans les îles Éparses et jusqu'en Méditerranée. Menaces de la faiblesse, celle des États faillis, qui nourrissent le terrorisme djihadiste. Menaces hybrides, créant des situations « troubles », dans la zone grise entre guerre et paix, l'utilisation de milices ou la désinformation massive. Nouveaux espaces de conflictualité : face au cyberespace, il faut aussi désormais l'espace extra-atmosphérique. De l'autre côté, les outils de régulation des crises internationales issus de la Seconde Guerre mondiale sont contestés : le Conseil de sécurité de l'ONU est bloqué sur la Syrie, sur le Yémen, sur le conflit israélo-palestinien. Le droit international est bafoué, la liberté de circulation des mers est contestée, les traités de maîtrise de la prolifération chimique et nucléaire sont fragilisés. Nos alliances les plus solides, comme la relation transatlantique, vacillent. L'Europe elle-même est frappée en plein coeur par la montée des populismes et la sortie de sa troisième puissance économique, le Royaume-Uni. Pourquoi, dans ce contexte, les crédits du Quai d'Orsay sont-ils si importants ? Parce que la France a, par sa diplomatie universelle, un rôle particulier à jouer sur la scène internationale. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, puissance militaire parmi les seules au monde à se projeter au-delà de ses frontières, nation qui « parle à tous », indépendante, dotée d'armées disposant d'une autonomie stratégique basée sur une capacité d'appréciation propre, la France est l'une des seules puissances mondiales à ne pas avoir « d'agenda caché » dans la gestion des crises. La France, pour résumer, ne vise qu'à « produire de la sécurité » et à se battre pour la paix.

Nous l'avons indiqué précédemment, l'aide au développement ne nous semble pas assez fermement pilotée du point de vue des priorités politiques. Nous l'avons dit samedi, notre notre confiance dans la bonne exécution de la loi de programmation militaire est désormais entamée : la défense a dû financer 400 millions de surcoûts des OPEX, qui auraient dû être pris sur la solidarité interministérielle. Venons-en à la diplomatie. Sur plusieurs sujets, la France n'est pas toujours au rendez-vous de son rôle historique. La vision un peu trop angélique qu'a l'exécutif du multilatéralisme ne nous permet pas de peser vraiment sur le cours des choses. Je déplore que nous soyons quasiment sortis des radars au Moyen-Orient, une région dont nous connaissons si bien les complexités. Il convient aussi de réinvestir l'Afrique, où notre est sévèrement contesté. Sur l'Europe, enfin, la vision très ambitieuse portée par le discours de la Sorbonne est quand même assez loin de la réalité. Prenons l'exemple du couple franco-allemand, qui- il faut bien le dire -ne pèse pas du même poids des deux côtés du Rhin

au « nouveau monde » qui a émergé, avec le Brésil, l'Inde, le Japon et des pays africains. Exactement ! Cette proposition joue aussi contre l'intérêt de l'Union européenne, qui est d'avoir plusieurs sièges au sein du Conseil de sécurité. J'espère que vous aurez l'occasion de le dire haut et fort à votre collègue allemand,

On se réjouit que les dépenses contraintes baissent ? C'est en fait le reflet de notre recul au classement économique international. Est-ce donc le moment d'amputer en plus cet outil d'influence qu'est le réseau diplomatique ? la réforme précipitée du Gouvernement est un non-sens. Pour économiser 110 millions d'euros, soit une demi-journée de dépenses de l'assurance maladie, on risque de se priver de leviers d'actions essentiels : amputer la diplomatie économique, alors que notre balance commerciale est décevante ; rogner sur l'action culturelle, alors qu'on lutte contre l'obscurantisme partout dans le monde

L'entretien lourd du patrimoine à l'étranger est doté de 12 millions d'euros, pour des besoins réels qui se situent entre 25 millions et 80 millions d'euros. Pis, la sécurisation de nos emprises à l'étranger n'est pas financée par des crédits budgétaires, mais par des cessions ! Car c'est bien à cela que mène le dispositif d'avance que Bercy vous a proposé pour 100 millions d'euros sur deux ans La commission le dit haut et fort : il faut mettre un terme à l'érosion du patrimoine qui découle de cette politique mortifère ! Monsieur le ministre, je veux vous donner acte que, depuis votre arrivée au ministère, cette politique a cessé.

qu'on les encourage et qu'on les aide à agir pour le bien et le rayonnement de la France et pour la paix. Très bien ! Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.

mais cela a un prix et nécessite un investissement. À ce titre, nous regrettons que la diplomatie économique soit considérée comme le levier majeur de notre diplomatie. Ce choix stratégique nous semble contestable. Il existe toujours malgré tout un reliquat de colonialisme dans notre pratique des échanges commerciaux avec certains pays, notamment d'Afrique. Ainsi, sous couvert d'aide au développement de ces pays, l'enjeu est aussi d'assurer un avenir international à nos entreprises. que le focus mis sur la diplomatie économique a conduit, par exemple, à une diplomatie politique des ventes d'armes, à propos desquelles vous connaissez notre opposition. Ces ventes massives d'armes n'ont pas développé d'emplois en France, puisque le secteur de l'industrie de l'armement a vu disparaître 44 000 emplois en dix ans. Dans le cadre de cette discussion budgétaire, je tiens aussi à intervenir sur un sujet

d'Afrique. Le maintien d'une zone franc après la décolonisation grève fondamentalement les capacités d'investissement des États et nuit à leur indépendance monétaire. Le franc CFA a le mérite de limiter l'inflation et d'apporter de la stabilité aux économies nationales, mais son indexation sur l'euro, une monnaie forte, freine de nombreuses PME africaines et encourage la fuite des capitaux.

de notre pays dans les pays concernés. Il faudra bien qu'on s'attelle un jour à ce problème. J'aborde maintenant un autre point : la nécessité de réinvestir massivement dans notre diplomatie culturelle. La situation de la diplomatie culturelle aujourd'hui est très délicate. C'est le domaine d'action qui présente le plus gros déficit entre les moyens mis en oeuvre et les besoins auxquels ils sont censés répondre. À ce titre, monsieur le ministre,

Cette ambition se fracture également avec l'exemple des étudiants étrangers. On ne peut que condamner la décision du Gouvernement d'augmenter drastiquement les frais d'inscription des étudiants étrangers à l'université. Dire qu'il s'agit d'une mesure visant à compenser ce que ces étudiants coûtent, c'est remettre en cause le sens même d'un service public Certes le principe du service public repose sur le caractère contributif de son fonctionnement, mais un étudiant étranger crée lui aussi de la richesse puisque, en travaillant, il consomme et paie des impôts indirects. Avec cette décision, vous ôtez tout espoir aux étudiants modestes de venir étudier en France, alors même qu'il existe déjà une barrière à l'entrée par le biais des revenus minimaux exigés.

Au-delà de leur accessibilité directe, cela empêche chaque année un certain nombre de jeunes étrangers de postuler dans l'une de nos universités. Alors que la France est le quatrième pays d'accueil d'étudiants étrangers, cette situation risque d'entraîner un recul de notre pays en la matière. Je terminerai en évoquant l'un des piliers les plus importants de notre action extérieure : notre réseau consulaire. La baisse des effectifs au sein des représentations françaises à l'étranger inquiète. Alors que le Quai d'Orsay a perdu 53 % de ses effectifs en trente et un tiers depuis 2008, le Gouvernement a encore annoncé la suppression de 10 % des effectifs. Aujourd'hui, on décompte seulement 13 800 agents pour 2 millions d'expatriés, sans tenir compte des touristes. J'y reviendrai lors de l'examen des amendements, mais le schéma « fermeture des accueils et dématérialisation des procédures » conduit à un certain recul.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'action extérieure de l'État, on le sait, est l'un des principaux instruments du rayonnement de la France dans le monde. À ce titre, il est important de préserver les moyens de la mission que nous examinons, ce maintien étant le gage de la diffusion des valeurs universelles qui nous sont chères. Avec une dotation de 2,9 milliards d'euros pour 2019 en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, j'observe, à périmètre constant, une diminution de 2,2 % des crédits par rapport à 2018.

puisque les dépenses de sécurisation des implantations à l'étranger relèvent d'un programme extérieur à la présente mission. Dans un monde multipolaire fragilisé, d'un côté, par la faiblesse des États faillis et, de l'autre, par les nouvelles stratégies de puissance, le projet kantien de paix perpétuelle demeure un idéal. Aussi, nous avons besoin d'un outil diplomatique efficace pour conserver à la France ses capacités d'influence et de pleine participation à la résolution des conflits. Cette influence, nous devons continuer à la déployer sur tous les fronts de l'action extérieure, que ce soit celui de la diplomatie culturelle, celui de notre emprise consulaire et, bien sûr, celui de notre implication dans les grandes organisations internationales. S'agissant de la diffusion de notre culture, la promotion de la langue française reste une composante majeure de notre diplomatie. Je me félicite donc de la sanctuarisation des crédits du programme 185. Toutefois, sans un soutien plus affirmé, il me semble que l'objectif de 700 millions de locuteurs au milieu de ce siècle, au lieu de 274 millions aujourd'hui, sera difficile à atteindre. Dans ces conditions, l'effort en direction du réseau des lycées français à l'étranger doit être conforté. N'hésitons pas aussi à nous appuyer davantage sur nos outre-mer pour mieux diffuser la francophonie. Pour ce qui concerne le réseau consulaire, je m'inquiète des conséquences que pourrait avoir la poursuite à marche forcée de la rationalisation qui affecte le programme 105. Je pense, en particulier, à la réduction de la masse salariale

je ne conteste pas le chantier de la mutualisation des fonctions supports de l'ensemble des ministères et opérateurs de l'État à l'étranger opéré dans le cadre du plan Action publique 2022. Je partage l'idée que cela contribuera à faire de chaque ambassade une véritable agence de l'État. Mais attention à ne pas effectuer ces réformes dans la brutalité, au risque d'affaiblir un réseau

au-delà du maillage des continents par nos ambassades, nos lycées et nos alliances françaises, c'est également au sein des grandes organisations internationales que la France expose son point de vue pour répondre aux défis du monde actuel.

l'a rappelé -que la France abandonne son siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations unies au profit de l'Europe. Or rappelons à nos amis Allemands qu'il faudrait au préalable que l'Union européenne ait une politique étrangère unique pour qu'elle ait un siège unique. Nous n'en sommes pas là ! J'ajouterai que ce n'est pas forcément avec des excédents budgétaires exemplaires que l'on répond aux défis stratégiques ... L'engagement des militaires sur les théâtres extérieurs est parmi les plus importants, ce qui justifie la place centrale de la France dans les instances multilatérales et sa légitimité à parler à tous. Sans prétendre à l'arrogance, nous devons préserver la place qui est la nôtre, car, au-delà de l'attractivité de notre pays, il s'agit de lui conserver son autonomie. J'entends bien sûr par autonomie celle qui nous permet de contrôler nos intérêts tout en continuant à nous ouvrir au monde, comme l'a très justement rappelé le Président de la République au Forum de la paix. de la paix. Le cycle mémoriel de la Grande Guerre, qui vient de s'achever, a ouvert des instants de commémoration rappelant que la paix d'hier avait été chèrement payée, et que celle d'aujourd'hui n'était pas éternellement acquise. ! Je vous encourage donc, monsieur le ministre, à poursuivre dans la voie de la consolidation de tous les outils diplomatiques qui se mettent au service des libertés humaines. Malgré tout, le groupe du RDSE votera ce budget.

Dans un contexte international dégradé, dangereux, instable, comme le montrent une fois encore les conditions du G20 ce week-end, le monde a besoin de plus de diplomatie et de plus de dialogue.

promouvoir farouchement le multilatéralisme. L'actualité internationale lui donne chaque jour un peu plus raison. Tout à fait ! Avec le troisième réseau diplomatique et consulaire, avec l'un des meilleurs corps diplomatiques au monde, avec des relais d'influence culturels, stratégiques et politiques anciens sur tous les continents, la France a toutes les cartes en main pour demeurer une grande puissance de diplomatie et de paix. Néanmoins, nous devons veiller à ne pas prendre pour acquise cette position unique sur la scène internationale. L'histoire nous montre que, lorsque nous cessons d'investir dans notre diplomatie et notre action extérieure, notre connaissance du monde s'amoindrit, notre voix s'affaiblit. À ce titre, l'affaiblissement continu du Quai d'Orsay et des réseaux culturels français depuis plusieurs années est inquiétant. II faut cesser de considérer notre action extérieure comme une variable d'ajustement. De l'aveu même de nombreux diplomates, le Quai d'Orsay est aujourd'hui à l'os. Je le dis aujourd'hui avec force : notre diplomatie est un actif précieux pour la France et un atout pour l'avenir Or vous semblez, monsieur le ministre, poursuivre dans cette logique de rabot progressif sur les crédits dédiés à cette mission, une fois corrigées les mesures de périmètre. Si nous croyons souhaitable la rationalisation du système de prime des agents diplomatiques, si des économies de fonctionnement sont encore possibles, nous estimons que la logique d'économies structurelles arrive à son terme, à moins de revoir drastiquement notre stature diplomatique. Cette stature, pour l'avenir, doit reposer sur trois piliers

D'autres pays affichent des efforts colossaux dans ce domaine : la Chine, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, par exemple, investissent massivement dans leur réseau culturel à l'étranger et occupent les espaces que nous délaissons. Notre propre réseau, atomisé et en perte de puissance, gagnerait à être rationalisé pour répondre à ce défi. Il pourrait s'appuyer sur une ambition renouvelée.

Face au retrait des États-Unis, face aux blocages persistants de la Russie, la France a une responsabilité accrue pour maintenir vivantes et efficaces les enceintes du multilatéralisme. Le troisième pilier est l'Europe. Elle est l'horizon naturel de notre action extérieure qu'elle a vocation à amplifier et à catalyser. Nous devrons oeuvrer à la construction d'une véritable politique extérieure commune- nous en parlons depuis tellement d'années ! -sur les grands sujets qui touchent à notre sécurité commune, aux crises dans notre voisinage et aux biens communs de l'humanité. Monsieur le ministre, ces points de vigilance ayant été rappelés, le groupe Les Indépendants-République et Territoires s'abstiendra sur ces crédits qui ne nous semblent pas à la hauteur des enjeux que doit affronter notre diplomatie.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la disproportion entre l'ampleur des efforts réclamés au Quai d'Orsay et son poids de moins de 2 % dans le budget de l'État est flagrante. Pour l'année prochaine, il lui est demandé de contribuer à 8 % de la baisse totale des emplois de l'État, alors qu'il ne représente que 0,7 % de l'ensemble de ses emplois Alors qu'il a déjà perdu 12 % de ses effectifs au cours de la dernière décennie, il reçoit cette fois l'injonction de conduire d'ici à 2022 une réduction de 10 % de la masse salariale de l'ensemble des réseaux français à l'étranger. Bien sûr, les Français de l'étranger ont un pouvoir de blocage limité, très inférieur à celui des gilets jaunes. Bien sûr, la saignée que l'on fait subir à nos ambassades et à nos réseaux culturels et économiques à l'étranger ne laisse que peu de traces visibles sur le sol français dans l'immédiat. Mais c'est là faire preuve d'une bien courte vue de la part du Gouvernement. Cynisme de Bercy ou bien réelle absence de vision à long terme ? Comment ne pas être exaspéré par le décalage entre les ambitions affichées et des moyens toujours plus restreints ? Oui nous devons, dans tous les domaines, apprendre à faire mieux avec moins Mais malgré l'immense qualité et le dévouement hors norme du personnel consulaire et diplomatique, auquel je tiens à rendre hommage, il faut cependant une baisse budgétaire minimale incompressible. Une réduction de 31 ETP pour le personnel consulaire ne permet pas de faire de vrais miracles. Ce budget pose aussi un problème de sincérité. Plusieurs des évolutions affichées s'apparentent à des tours de passe-passe. C'est notamment vrai pour notre patrimoine immobilier à l'étranger. Notre histoire nous a légué de véritables joyaux qui constituent une véritable vitrine de la France à l'étranger : si une gestion innovante est nécessaire pour mieux en optimiser l'usage, gardons-nous de les brader, surtout dans des conditions de transparence douteuses. Je note aussi que 30 millions d'euros non inscrits au budget seront consacrés en 2019 et en 2020 à des investissements de sécurité dans le réseau sous forme d'avances, avances que le ministère devra rendre entre 2021 et 2025 par des cessions de biens immobiliers. Je soutiens donc la proposition, qui n'est pas si baroque que cela, de notre collègue Robert del Picchia de les vendre à des institutions françaises, comme la et consignations. De même, la suppression de la réserve parlementaire s'est traduite par une perte nette de budget pour nombre de structures françaises à l'étranger. Non seulement le dispositif STAFE, censé la remplacer, est bien moins doté d'un tiers, mais il décourage de nombreuses petites associations, incapables de trouver elles-mêmes la même somme en autofinancement. Plus inquiétant encore, nous assistons à des effets de substitution où des budgets dépendant autrefois de l'action extérieure de l'État passent désormais sur la ligne STAFE. Je l'ai noté à Londres justement. Le nombre de Français à l'étranger ne cesse d'augmenter, et les moyens ne suivent pas. Soyons bien conscients qu'une stagnation des budgets équivaut, sur le terrain, à une dégradation des services publics. Le budget des bourses scolaires, par exemple, va continuer de baisser : il sera cette année amputé de 5 millions d'euros. Cela fait des années que nous demandons une étude sérieuse sur l'effet conjugué de l'augmentation des frais de scolarité de la réforme du système de bourses. Malgré les dénégations des gouvernements Hollande et Macron, il est clair que les classes moyennes et les familles à faible revenu sont en train d'être écartées de nos écoles. L'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger subira une diminution de 3,7 % de ses crédits et une baisse de 166 équivalents temps plein. Ces nouvelles contraintes sont imposées alors même que les effectifs d'élèves ne cessent de croître, occasionnant des dépenses en hausse. Emmanuel Macron s'est même engagé à doubler le nombre d'élèves scolarisés dans nos écoles françaises à l'étranger. Cherchez l'erreur ! Ce sont évidemment les frais de scolarité qui vont flamber. Alors que le Président de la République a multiplié les annonces en faveur de la francophonie, ce dont nous lui sommes reconnaissants, les crédits du programme « Diplomatie culturelle et d'influence » baisseront de 2,6 %, après une année 2018 stable et deux années de recul. La faible augmentation des crédits aux instituts français et alliances françaises n'est pas pas à la hauteur des enjeux. Au-delà des questions budgétaires, les modalités du rapprochement de ces deux réseaux demeurent floues et laissent craindre des fermetures de centres culturels, de vastes zones, voire des pays entiers, risquant de se retrouver sans foyer de diffusion francophone. Ce budget pour 2019 donne l'impression que le Quai d'Orsay, déjà affecté par des années de rabot budgétaire, est maintenant à l'os et en est réduit à des expédients et à des économies « de bouts de chandelles ». Je ne reviendrai pas ici sur la menace de suppression des journées défense et citoyenneté à l'étranger,

supprimant les JDC nous refusons la diffusion de nos valeurs parmi nos jeunes compatriotes et binationaux à l'étranger. À un moment où cela est indispensable, nous nous privons de nos meilleurs ambassadeurs de demain. Ce serait une faute aussi morale que stratégique La France a toujours eu une place à part dans les relations internationales. Dans ce village global où les rivalités font rage, nos concurrents ont, eux, bien compris que le progrès et le développement économique passaient obligatoirement par l'international. Ils se donnent, eux, les moyens de leur réussite. Dans quelques années, nous risquons de regretter notre aveuglement si nous ne prenons pas les mesures adéquates. La

consulaires sont à la tâche aux quatre coins de la planète. Ils ont cette mission impérieuse de nouer, de tisser et de maintenir des relations entre notre pays et le reste du monde. Ils ont aussi cette lourde responsabilité de s'adapter à la croissance continue de nos communautés à l'étranger et de les protéger. Je voudrais leur rendre hommage, les remercier, au nom de la représentation nationale, pour leur travail au service de la France, pour leur engagement immuable, pour leur immense impact dans tous les coins et recoins du monde. Ils font face à de multiples défis, l'environnement stratégique mondial étant durablement marqué par l'incertitude et l'instabilité. Je pense ainsi au changement climatique. La COP24, qui s'est ouverte hier en Pologne, comme les signes déjà visibles des dérèglements climatiques sont là pour nous rappeler l'urgence d'agir ensemble, l'urgence de trouver des solutions ambitieuses pour sauver notre planète et pour nous assurer que, demain, nos enfants et nos petits-enfants ne naîtront pas condamnés. Je pense aux défis sécuritaires, qui engagent nos intérêts et nos forces civiles et militaires, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Je pense aux grands mouvements migratoires, aux remises en cause du libre-échange et de la stabilité de l'ordre international ou encore aux coups portés au projet européen. Pour compliquer encore la donne internationale, tout comme nos actions diplomatiques, le multilatéralisme hérité du siècle passé est aujourd'hui sérieusement ébranlé. Des puissances comme les États-Unis, qui, hier encore, défendaient ce système, se mettent désormais à le contester, préférant jeter leur dévolu sur un repli nationaliste bien plus qu'inquiétant. Nous ne pouvons que le regretter amèrement. Toutes ces questions sont prépondérantes pour notre diplomatie. Elles sont cruciales pour notre avenir. C'est pourquoi notre pays doit pouvoir continuer à compter sur un outil diplomatique efficace et crédible. Avec un budget de 2,79 milliards d'euros dédié à la mission « Action extérieure de l'État », le ministère de l'Europe et des affaires étrangères subit une diminution d'environ 4 %. Comme vous aviez eu l'occasion de l'expliquer, monsieur le ministre, cette baisse s'explique à la fois par une réduction du coût des contributions internationales et des opérations de maintien de la paix, par une diminution de la quote-part française et par une gestion améliorée du risque de change par votre ministère. Ce montant est aussi à mettre en perspective avec le budget global du Quai d'Orsay, d'un montant de 4,89 milliards d'euros, mission « Aide publique au développement » comprise. Au total, le ministère bénéficie d'une hausse de plus de 151 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2018. Cette hausse, répercutée dans l'aide publique au développement, est inégalée et salutaire, puisqu'elle est un précieux outil de l'influence internationale de la France. Elle nous permet d'adopter une approche globale et concrète des crises et des enjeux internationaux. Avant tout, le budget de la mission « Action extérieure de l'État » reflète notre fervent engagement envers le multilatéralisme et la sécurité collective, ainsi qu'envers les acteurs qui l'animent et agissent au quotidien pour rendre le monde plus équitable et moins incertain. Le maintien de notre rang international est porté par cet engagement. Il passe par notre participation et nos contributions obligatoires aux opérations de maintien de la paix conduites sous l'égide de l'ONU, qui atteignent 326 millions d'euros. Il passe aussi par notre action constante au sein des organisations internationales. Notre contribution à leur fonctionnement s'élève à 194 millions d'euros en crédits de paiement pour 2019. Concrètement, cet argent servira à soutenir le travail remarquable effectué par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en faveur de l'action humanitaire ou encore celui mené par l'UNICEF pour les droits des enfants. enfants. Ce budget est aussi celui du renforcement de l'influence et de l'attractivité de la France dans le monde. Étant donné l'importance des ambitions de renforcement de notre attractivité universitaire et de diffusion de notre culture et de notre langue, nous nous réjouissons de la sanctuarisation des moyens de notre réseau de coopération et d'action culturelle, comme vous l'aviez promis l'an passé, monsieur le ministre, au moment d'acter une hausse de ce budget, dans la loi de finances pour 2018. Ainsi, les crédits alloués à l'Institut français sont rehaussés, après avoir diminué de 11 % entre 2012 et 2017, ... C'est artificiel ! ... tandis que les bourses d'étudiant sont sanctuarisées. Soulignons que notre réseau d'enseignement français est unique au monde et scolarise 350 000 élèves dans 500 établissements. De même, notre groupe tient à réaffirmer son soutien pour le travail exceptionnel et complémentaire qu'effectuent le réseau des Instituts français et celui des Alliances françaises. Enfin, ce budget doit permettre d'acter une réforme structurelle du ministère, attendue de longue date, qui s'inscrit dans le cadre de la démarche de modernisation Action publique 2022. Le Quai d'Orsay se voit effectivement confier le pilotage de l'ensemble des réseaux de l'État à l'étranger. L'ambassadeur en poste devient le chef de file de l'ensemble de son équipe. Il aura une vision globale sur les moyens dont il dispose et fixera les compétences requises au regard du plan d'action de l'ambassade. Nous nous félicitons de cette unité budgétaire et de commandement, qui aura un impact positif direct sur la qualité de nos actions diplomatiques. Elle permettra à notre diplomatie de mieux embrasser les priorités thématiques et géographiques. À travers ses 163 ambassades, la France a la responsabilité de faire entendre sa voix au nom de la paix, de la prospérité mondiale et du bien commun. Face à cette tâche immense qui nous incombe, nous savons, monsieur le ministre, que nous pouvons compter sur votre engagement total, ainsi que sur celui du Gouvernement. Le groupe La République En Marche votera par conséquent en faveur des crédits de la mission « Action extérieure de l'État », pour témoigner de son soutien en faveur de notre diplomatie.

Nous en avons plus que jamais besoin ! Notre pouvoir d'influence à l'international reste fort, parce que nous avons fait le choix, fruit d'une longue tradition, d'être présents physiquement grâce à notre réseau diplomatique et consulaire, considéré comme l'un des premiers au monde, et grâce à notre présence culturelle éducative et économique. La France compte ! On nous fait confiance, parce que nous allons au contact porter notre voix, et vous êtes le premier à montrer l'exemple. C'est bien notre force de persuasion et d'attraction qui a fait de la COP21 un formidable succès pour notre pays. Pourtant, notre diplomatie souffre d'une vision obsolète du rôle de l'ambassadeur, se traduisant par des choix budgétaires qui ne sont guère en faveur du Quai d'Orsay, traité depuis longtemps par le ministère des finances comme une variable d'ajustement. Cela se traduit, notamment, par la vente et le retrait de nos antennes et de certaines missions à l'étranger, qui entraînent immédiatement une baisse de la présence française, toujours très mal perçue par nos ressortissants et les autorités des pays concernés. Si vous vous inscrivez dans un mouvement qui n'est pas nouveau, son ampleur est nouvelle. Vous nous annoncez une ponction inédite de 10 % sur la masse salariale de toutes les missions, ce qui entraînera d'importantes suppressions de postes. Vous en conviendrez, on nous impose un vrai massacre à la calculette. Les effectifs concernés, 130 pour 2019, sont issus de plusieurs ministères. Néanmoins, six de vos collègues du Gouvernement, et non des moindres- les ministres de l'action et des comptes publics, de l'économie et des finances, de l'agriculture, des armées, de l'intérieur et de la transition écologique ont d'ores et déjà annoncé qu'ils refusaient de se laisser imposer de futures suppressions de postes internationaux par votre ministère. Allez-vous être forcé de concentrer ces économies sur le seul Quai d'Orsay ? ? Si vous deviez supporter majoritairement les suppressions demandées, celles-ci entraîneraient indéniablement la fermeture de nombreuses ambassades et consulats et mettraient fin, d'un coup, à ce que nous avons laborieusement construit depuis longtemps. Cela nous amènerait également à entamer de longues négociations pour payer des primes de licenciement à des personnels recrutés localement, qui ont souvent fait toute leur carrière au service de la France. Les économies réalisées risquent fort de nous coûter très cher sur le long terme. L'image de la France sera également ternie. Dans ce contexte, pourriez-vous préciser quelles sont les intentions du ministère de l'Europe et des affaires étrangères quant à cette politique de suppressions de postes ? J'imagine que la dématérialisation et l'externalisation seront accélérées, alors qu'elles ne sont pas accessibles par tous et partout. Je regrette le choix d'un service public d'où disparaît progressivement le contact humain, pour des raisons comptables. Heureusement, nous avons nos 442 conseillers consulaires, qui sont nos meilleurs liens de proximité avec les Français établis hors de France et qui sont élus, notamment, pour les conseiller et les accompagner lors de leurs démarches administratives.

Nous avons 497 établissements implantés dans 197 pays, gérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; 350 000 élèves y sont scolarisés, avec une augmentation de 2 % par an de ces effectifs. Après l'annulation de 33 millions d'euros des crédits de l'AEFE en 2017, le taux de participation financière complémentaire versée par les établissements conventionnés est passé de 6 points à 9 points en 2018 pour compenser cette baisse. Ce sont les familles qui ont été mises à contribution, avec une augmentation des frais de scolarité. Il n'est pas logique de conserver une enveloppe des bourses à budget constant, alors que la demande croît, de par l'augmentation des frais de scolarité et de par la hausse de 3 % par an de nos communautés françaises présentes à l'étranger. Le Président de la République a annoncé vouloir doubler le nombre d'apprenants de français dans le monde. Nous avons donc besoin de davantage d'établissements pour les accueillir, nécessitant plus de moyens financiers et humains. Or la décision d'arrêter brutalement la garantie de l'État, accordée jusqu'alors par l'Association nationale des écoles françaises de l'étranger, l'ANEFE, bloque aujourd'hui l'agrandissement de certains établissements et ne permettra pas à d'autres de contracter les prêts nécessaires. Un remplacement de ce système de garantie est-il recherché afin de sortir ces établissements de l'impasse dans laquelle ils se trouvent et qui engage leur stabilité financière et l'avenir scolaire des élèves qui y sont scolarisés ? Ce retrait de l'État est-il la première étape vers la recherche d'investisseurs privés qui se substitueront à lui ? Si le doublement du nombre d'élèves semble reporté à 2030 dans les documents budgétaires du projet de loi de de l'engagement présidentiel d'origine, cet objectif ne pourra être atteint que si le recrutement des professeurs, et surtout leur détachement, est planifié. Or la réduction du nombre des enseignants, après cinq ans d'augmentation, et la circulaire limitant leur détachement ne vont pas dans le sens de la hausse importante du nombre de détachements dont le réseau aura besoin. Sans compter les postes nécessaires au réseau de la Mission laïque française, conseillers culturels, directeurs d'alliances françaises et d'instituts français. L'ambition constante du Président de la République à déployer une diplomatie universelle et des services consulaires de qualité pour nos compatriotes établis hors de France est incompatible avec son engagement de réduire, en même temps et dès 2019, le budget du ministère sur ces missions essentielles à notre service public. C'est l'image et le rayonnement de la France qui sont en jeu, partout dans le monde. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'examen de la mission « Action extérieure de l'État » que nous abordons aujourd'hui est un rendez-vous essentiel pour la vie des Français vivant hors de nos frontières, ces compatriotes que j'ai l'honneur de représenter au sein de cette assemblée. Avant de commencer mon intervention, je souhaite témoigner que l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République a donné un lustre à l'image de notre pays à l'international que nous n'avions pas connu depuis très longtemps. C'est une source de satisfaction pour tous ceux qui sont attachés à promouvoir la France à l'étranger. Pourvu que ça dure En quatre ans de mandat, j'ai effectué 289 déplacements dans 79 pays à l'étranger. Cela m'a permis d'engager un contact étroit avec nos ambassadeurs, nos conseillers consulaires, qui forment le tissu de nos élus locaux à l'étranger, nos consuls, nos consuls honoraires honoraires et tous les acteurs des domaines économique et culturel. Je souhaite ici tous les remercier pour leur aide et leurs suggestions afin de m'aider dans mes missions.

Je tiens à ce titre à saluer nos rapporteurs, notamment mes collègues de l'Union Centriste Claude Kern et Vincent Delahaye, pour la qualité de tous leurs travaux dans ces domaines. ces domaines. La baisse globale des crédits dédiés à l'action extérieure de l'État va dans le sens souhaité par les Français d'une réduction de la dépense publique. si nous pouvons être d'accord sur l'objectif, nous émettons des réserves sur les chemins empruntés pour y parvenir. Comme certains l'ont dit, pour le Quai d'Orsay, Bercy a inventé le coup de rabot permanent. Commençons par la réduction moyenne de la masse salariale de 10 % d'ici à 2022. La méthode engagée pour y parvenir a des effets qui conduisent les personnels en poste au découragement. Pour obtenir l'adhésion, il faudrait assortir cette démarche d'une vision qui permette aux 90 % des agents restants de s'attendre à ce que leur futur soit plus glorieux. Nos ambassades, nos résidences sont la vitrine de la France à l'étranger ! C'est ce qui nous permet de communiquer. J'ai pu constater à Hong Kong ou Cape Town que la vente de nos résidences pour financer l'entretien d'autres biens dégradait notre image localement.

Nous n'avons plus beaucoup de marges de manoeuvre. M. Gourdault-Montagne a rappelé que notre immobilier n'était financé que par des cessions, et ce qu'il s'agisse de maintenance ou de construction. Depuis une dizaine d'années, nous avons donc débudgétisé l'immobilier. Nous avons connu, en 2018, onze opérations de cession à l'étranger, pour un total de 30 millions d'euros. Nous aurons, en 2019, un montant à peu près équivalent, ce qui n'est pas suffisant et a entraîné, par exemple, la suspension de la construction d'une nouvelle ambassade en Corée. n'investissons pas suffisamment dans l'entretien de nos bâtiments, ils se dégradent. Déjà, l'an dernier, nous vous posions ici la question suivante, restée sans réponse : quelle est, monsieur le ministre, la stratégie du Gouvernement à moyen terme dans ce domaine ? Dans le cadre de la « modernisation des services consulaires », nous proposons en outre plusieurs pistes de travail qui servent toutes cette ambition d'offrir un service public de qualité aux Français de l'étranger. Nous avons de plus en plus d'expatriés, mais de moins en moins de moyens, c'est le fameux effet ciseaux. Nous souhaiterions expérimenter une approche plus audacieuse, au terme de laquelle les consulats seraient transformés en centres de profit la récupération intégrale du produit des services fournis. Parmi les solutions envisagées pourrait figurer également l'équipement d'outils de saisie d'empreintes biométriques pour les consuls honoraires, à l'image de ce que font nos amis Allemands. Autre sujet majeur : l'enseignement français à l'étranger. Tout d'abord, je veux faire Je vous proposais à cette tribune l'an dernier, au nom du groupe Union Centriste, l'objectif de doubler le nombre d'écoles françaises à l'étranger d'ici à cinq ans.

Je me félicite que le réseau se mette « en marche », même si je regrette que cela soit une marche lente. Nous espérons que cela aboutira à une profonde réforme de l'AEFE, et nous nous réjouissons que le Premier ministre ait confié une mission à la députée Samantha Cazebonne Nous appelons de nos voeux une transparence totale sur les dépenses de l'AEFE, qui, je le rappelle, n'accueille qu'un enfant français sur cinq établis à l'étranger.

ne trouvez-vous pas, monsieur le ministre ? Enfin, la politique de coopération culturelle constitue une part essentielle de l'action de la France à l'étranger. Elle permet à notre pays de rayonner hors de ses frontières auprès de publics étrangers, tout en s'adressant aussi à nos compatriotes expatriés. Nous saluons donc la hausse du budget alloué à ces actions dans le programme 185, bien que nous en déplorions la faiblesse des montants. Pour quatre enfants français sur cinq à l'étranger, les familles doivent donc se tourner vers l'enseignement local, voire vers les établissements internationaux. De fait, de nombreux enfants nés de couples binationaux ne parlent aujourd'hui pas notre langue, et ce alors même qu'ils disposent de la nationalité française. L'objectif que nous proposons, comme nous l'avions fait l'an dernier, est que tous les Français parlent français. Je soumettrai donc trois amendements visant à apporter une réponse à cette problématique par le transfert des crédits de l'AEFE vers l'Institut français, pour financer l'expérimentation d'un chèque éducation ouvert à tous les enfants français à l'étranger. Cela participera au financement de l'Institut français et des alliances françaises, qui réalisent un travail essentiel de diffusion de la langue et de la culture françaises hors de nos frontières. Dans un contexte de stagnation budgétaire, nous nous félicitons que l'Institut français fasse figure d'exception, puisque sa subvention augmente de près de 7 %. De même, les subventions aux alliances françaises croissent de 6 % pour mettre en oeuvre le plan en faveur de la langue française. Or la Fondation Alliance française reste dans une situation difficile. Mon groupe aura donc l'occasion de vous soumettre un amendement visant à la soutenir.

Je salue d'ailleurs l'annonce de la future loi de programmation énergétique. La mission « Action extérieure de l'État » est essentielle à l'heure de la redistribution des positions et des mutations géostratégiques, dans un contexte où les moyens d'influence se complexifient et se multiplient. Nous devons surtout ne pas oublier que les luttes d'influence ne sont plus seulement le fait d'États et de groupes politico-militaires, mais également de géants économiques.

je souhaite souligner la qualité et la richesse des travaux de la commission, sous la présidence de Christian Cambon. J'espère, monsieur le ministre, que vous ne serez pas sourd aux observations que nous avons formulées

le budget de la mission « Action extérieure de l'État » est reconduit à périmètre constant. J'y insiste, toutes les dotations de cette mission sont reconduites à périmètre constant.

de la décision de conforter le ministère de l'Europe et des affaires étrangères dans son rôle de pilotage interministériel de l'ensemble de l'action extérieure de l'État. J'ai fait précédemment référence à la partie immobilière. Il s'agit de créer une véritable agence de l'État à l'étranger, sous l'autorité de l'ambassadeur. Désormais, la gestion des fonctions supports et des crédits de fonctionnement de tous les réseaux internationaux de l'État, aujourd'hui disséminés, sera unifiée sous la seule responsabilité du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. C'est une mutation considérable, et je remercie les rapporteurs spéciaux d'avoir bien voulu à l'effet « silo » de la gestion des moyens de l'État à l'étranger. Il est vrai qu'en contrepartie de ces réorganisations et dans le cadre de la maîtrise des dépenses de l'État, le Premier ministre a fixé un objectif

Ce projet de budget doit nous permettre de mettre en oeuvre les grandes priorités de notre diplomatie. La première d'entre elles est le soutien au multilatéralisme et, plus largement, aux acteurs

se produire alors. La deuxième priorité assignée à mon ministère est de renforcer l'influence et l'attractivité de notre pays. C'est pourquoi j'ai souhaité que les moyens de notre réseau de coopération et d'action culturelle soient sanctuarisés.

à l'étranger seront maintenus, conformément aux engagements du Président de la République. L'AEFE recevra ainsi une subvention de 384 millions d'euros. Le modèle de l'Agence sera conforté, et nous engagerons

à 105 millions d'euros vise simplement à adapter le budget à la dépense réelle observée. Je tiens d'ailleurs à vous préciser que, lors de la discussion budgétaire en séance publique à l'Assemblée nationale, en réponse à plusieurs amendements déposés sur la possibilité d'augmenter le nombre de familles bénéficiaires d'une aide à la scolarité, j'ai annoncé que j'allais étudier la revalorisation du barème du quotient familial maximum de 21 000 à 23 000 euros pour la rentrée 2019-2020. Cette mesure n'est pas d'ordre législatif, mais je

enfin les opérateurs, l'accroissement des moyens de l'Institut français, à hauteur de 2 millions d'euros, permettra notamment de financer les actions liées au plan Francophonie annoncé par le Président de la République en mars dernier.

poursuivre notre vigilance sur la bonne qualité de la mobilisation des fonds qui y sont affectés. À cet égard, je voudrais rassurer M. Cadic : notre ambassade à Séoul sera la première priorité de notre programmation en 2019. Je sais qu'il y a

ce programme a été paramétré pour faire face aux besoins les plus indispensables, et guère plus. Nous avons une maîtrise très rigoureuse de ces crédits, sous le contrôle de la Cour des comptes. La vigilance sera donc totale. Tels sont les quelques propos complémentaires dont je voulais vous faire

les moyens mis à disposition me permettent d'agir et permettent à l'ensemble des acteurs du Quai d'Orsay d'agir de manière cohérente et efficace.

Ces amendements traitent de thématiques très variées. Malgré l'existence d'incompatibilités de fond, ils ont été inscrits en discussion commune, car, d'une part, deux d'entre eux visent à prélever des crédits sur l'action n° 05 du programme 185 pour un montant cumulé supérieur aux crédits inscrits et, d'autre part, huit d'entre eux tendent à prélever des crédits sur le programme 347 pour un montant cumulé très supérieur aux crédits inscrits. En conséquence, en cas d'adoption d'amendements,

faute de moyens. En se basant sur les deux tiers des agents qui « badgent », les heures écrêtées effectuées et les congés perdus représentent 70 emplois à temps plein. Il existe donc un vrai différentiel entre les besoins

expatriés. Entre une surcharge de travail pour les agents et la fermeture d'antennes locales consulaires, les Français à l'étranger sont de plus en plus nombreux à renoncer à certaines démarches administratives.

Cette dématérialisation peut effectivement constituer une alternative importante, à condition qu'elle ne remplace pas la possibilité de se déplacer- mais je ne développerai pas davantage.

le dernier tiers est constitué de contractuels intérimaires de droit français. Cette répartition revient évidemment beaucoup moins cher à l'État, puisque les rémunérations et les perspectives de carrière sont extrêmement limitées.

Cet amendement a pour objet de permettre le financement des actions en faveur de l'enseignement du français pour les élèves de nationalité française vivant à l'étranger. Les fonds ainsi transférés du programme 185 vers le programme 151 ont en effet vocation à être réinjectés deux autres amendements, que je présenterai dans quelques instants, dans le programme 185, et notamment son action n° 02 « Coopération culturelle et promotion du français

L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a subi, dans le projet de loi de finances rectificative pour 2017, une annulation de crédits d'un montant de 33 millions d'euros qui a placé ce réseau dans une position plus que délicate. Cette annulation de crédits a fragilisé l'AEFE, qui se trouvait déjà en situation de sous-financement depuis le transfert à l'Agence des compétences relatives au patrimoine immobilier ainsi que de la charge des pensions civiles,

nationale. Elle a également affaibli ses capacités d'intervention, d'investissement et sa capacité de pilotage, dans un réseau pourtant largement reconnu dans le monde et indispensable à notre diplomatie d'influence. Cette baisse de crédits survient alors que le Président de la République a fixé lui-même l'objectif de doubler le nombre d'élèves scolarisés à l'étranger d'ici à 2030. On ne peut énoncer un tel objectif ambitieux et, en même temps, ne pas se donner les moyens financiers de l'atteindre, surtout lorsque l'on constate une augmentation croissante des effectifs à un niveau de 2 % en moyenne par an. Il conviendrait, à l'inverse, que l'enseignement français à l'étranger et son opérateur public, l'AEFE, connaissent une augmentation de budget dans le cadre du projet de loi de finances pour

: La parole est à M. Damien Regnard. Cet amendement vise à augmenter de 4,7 millions d'euros la subvention pour charges de service public versée à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger afin de compenser, dans sa totalité, les effets de l'annulation d'une partie de la subvention en juillet 2017.

350 000 élèves sont scolarisés dans 492 établissements homologués à travers 137 pays. Le seuil de tolérance des familles est désormais atteint et le désengagement progressif de l'État devient menaçant.

à réduire d'autant les crédits de paiement de l'action « Préparation et organisation du sommet du G7 » au sein du programme « Présidence française du G7 ». Nous préférons flécher les crédits au bénéfice du plus grand nombre, même si nous souhaitons le plus grand succès du G7, puisque cet amendement vise à soutenir l'action de notre réseau des ambassades afin de préserver la sécurité des postes à l'étranger. L'amendement n° II-29 rectifié, présenté par MM. Regnard : La parole est à M. Damien Regnard. Cet amendement vise à soutenir le dispositif des bourses scolaires en faveur des familles à revenus modestes et à accompagner les élèves en situation de handicap. Les familles qui rencontrent des difficultés pour faire face aux frais de scolarité doivent pouvoir être soutenues et accompagnées afin que l'excellence des enseignements dispensés par les établissements du réseau de l'AEFE leur soit également accessible.

Le programme 151 affirme ainsi qu'il faut stabiliser la dotation annuelle consacrée à l'aide à la scolarité des enfants français inscrits dans les établissements du réseau de l'AEFE à son niveau de 110 millions d'euros. Or le programme prévoit une aide à la scolarité budgétée à 105 millions d'euros, auxquels s'ajouterait un prélèvement de 5 millions d'euros sur des liquidités accumulées au sein de l'AEFE. Cette soulte ne soulte ne peut être considérée comme un maintien au même niveau des dotations dédiées à l'AEFE ; elle relève plutôt de l'artifice comptable. Elle a été constituée au cours des années antérieures par des trop-perçus et des gains au change des années précédentes. Le Gouvernement affirme que l'AEFE disposerait des moyens nécessaires pour faire face au coût anticipé de la campagne des bourses et aux risques éventuels d'une perte au change ou d'une augmentation des frais de scolarité.

Or nous savons que l'AEFE ne dispose pas des moyens nécessaires pour faire face à cette augmentation de 5 millions d'euros. La diminution des dotations entraîne une augmentation des frais de scolarité, qui touche, de fait, les familles les plus modestes. Les demandes de bourses s'en trouvent ainsi augmentées, et toutes ne sont pas satisfaites à hauteur des besoins. La tendance est d'ailleurs à s'attaquer aux boursiers à 100 % en réduisant leur quotité pour des raisons budgétaires. De nombreux établissements doivent aussi faire face à de plus en plus d'impayés, en raison des difficultés financières des familles. De telles situations sont intolérables. Alors que le Président de la République souhaite doubler le nombre d'apprenants du français, faudra-t-il alors que ces lycées soient réservés aux plus privilégiés ?

Cette stratégie, censée améliorer notre capacité à attirer davantage d'étudiants et à faire face à la concurrence des pays étrangers, fait quasiment l'unanimité contre elle. Il est vrai que l'on peut s'interroger sur l'efficacité de cette stratégie, qui repose principalement sur l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Si je peux concéder que l'augmentation du prix des formations pourrait attirer certains étudiants de nationalité chinoise ou indienne, pour qui un prix élevé de scolarité est souvent synonyme de qualité, cette hausse va nécessairement nous priver d'étudiants plus modestes. En effet, le droit d'étudier sera désormais fixé à 2 770 euros en licence, contre 170 euros aujourd'hui, et à 3 770 euros en master et en doctorat, contre 243 euros en master et 380 euros en doctorat aujourd'hui, soit un prix prohibitif pour de nombreux étudiants. eux, notamment en Afrique francophone, ont réagi avec tristesse et colère à vos annonces. Ils ont en effet eu le sentiment d'être trahis. Comment ne pas les alors que le Président de la République avait indiqué à plusieurs reprises ces derniers mois son ambition pour la francophonie ? Au regard de cette stratégie, cette ambition francophone ne me semble plus crédible. Monsieur le ministre, au lieu d'augmenter les frais d'inscription, nous vous proposons, par cet amendement visant à renforcer le budget de Campus France de 5 millions d'euros, d'améliorer significativement l'accueil et les conditions de vie des étudiants étrangers.

Pour 2017, 3,34 millions d'euros de crédits étaient inscrits dans le projet de loi de finances au titre de la réserve parlementaire des députés et sénateurs des Français de l'étranger, au programme 151, « Français à l'étranger et affaires consulaires », dans la mission « Action extérieure de l'État Ces crédits budgétaires apportaient une contribution vitale à la vie associative française à l'étranger, que ce soit dans le domaine de la culture, de la solidarité ou de l'emploi. Pour compenser la suppression de la réserve parlementaire, prévue à l'article 14 de la loi organique n° 2017 1338 du 15 septembre 2017

Pour 2019, le programme 151 a été doté de 2 millions d'euros. Pourtant, le 2 octobre 2017, devant l'Assemblée des Français de l'étranger, le Président de la République a déclaré Je demande au ministre de l'Europe et des affaires étrangères [ ...] d'étudier la mise en place d'un dispositif permettant d'accompagner le tissu associatif des Français de l'étranger compte tenu de la suppression de cette réserve. Nous devons avoir là un principe de justice, je sais que pour beaucoup d'associations que vous souteniez et que les parlementaires accompagnaient, la réserve était un élément important et donc nous devons regarder là-dessus comment créer avec le Quai un dispositif comparable et que les ministres puissent instruire cela en lien avec vous-même et les parlementaires. » Or le STAFE est très loin de compenser la réserve parlementaire. Entre 2017 et 2019, l'effort budgétaire en direction des associations françaises à l'étranger a baissé de 40 %. De fait, l'immense majorité des associations françaises qui structurent le lien social des communautés à l'étranger sont abandonnées par l'État. elles remplissent une mission essentielle d'intérêt général et ne peuvent s'appuyer sur aucune autre personne publique, qu'il s'agisse du maire, du conseil départemental ou du conseil Le système d'« appel à projets » est inégalitaire, dans la mesure où il favorise les associations les plus importantes, lesquelles sont déjà les mieux positionnées pour lever des fonds. Il est aussi peu démocratique, car il exclut les parlementaires du processus de sélection des projets.

est en cours de règlement. Cet assainissement, qui va permettre de préserver une tête de réseau mondial, interface entre les sociétés civiles locales, dont les alliances sont l'émanation, et notre diplomatie d'influence, n'est toutefois pas

Avec moins de dix agents, elle court le risque d'être incapable de faire face à ses missions au service de quelque 835 alliances. Le présent amendement a donc pour objet de transférer 600 000 euros du programme 347

programme 185 et de ceux de l'AEFE. Sur la forme, la création d'un programme dédié à la promotion du français n'apparaît pas comme une nécessité en l'état de la maquette budgétaire.

Une telle hausse ne semble pas nécessaire, d'autant que nos travaux ont mis en évidence les chantiers de modernisation du réseau consulaire à moindres frais. L'avis est donc défavorable.

Pour 2019, Campus France devrait bénéficier de 81,3 millions d'euros de financement public, soit 16 % de plus qu'en 2016. Sa subvention pour charges de service public versée par la mission « Action extérieure de l'État » est stable entre 2018 et 2019, à 3,8 millions d'euros. Depuis 2016, l'attractivité de l'enseignement supérieur français pour les étudiants étrangers se confirme. Le nombre d'étudiants étrangers en mobilité en France est ainsi passé de 184 000

Selon les informations transmises par le ministère à vos rapporteurs spéciaux, il n'a démarré qu'à la moitié de l'année 2018, entraînant des retards dans l'instruction des dossiers. Toutefois, les postes diplomatiques et consulaires semblent s'être bien approprié cet outil, puisque, début octobre, 302 projets émanant de 112 postes diplomatiques avaient été reçus et examinés par la commission consultative du STAFE.

le Premier ministre a demandé à Mme Cazebonne d'établir un diagnostic sur la situation des effectifs scolarisés en français

parlementaire, c'est le G7 ... Au regard de l'objectif du Président de la République de doubler le nombre d'élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger, il est absolument impératif que tous ceux ayant fait leurs études dans nos établissements et qui sont titulaires du baccalauréat puissent bénéficier des mêmes tarifs qu'actuellement.

ministre, vous avez raison de signaler que le nombre d'étudiants étrangers a augmenté en France de 4,6 %. Mais, dans le monde, l'augmentation est de près de 7 %, en sorte que la France a perdu un rang, au profit de l'Australie, et en perdra sans doute deux autres l'année prochaine, au profit de la Russie

notre commission ne manque jamais de visiter les alliances françaises et les instituts français. Partout dans le monde, nous constatons un certain nombre de difficultés, d'autant que les moyens de la mission « Action extérieure de l'État », pour le volet « diplomatie culturelle », ont été considérablement réduits lors du précédent quinquennat, il faut le rappeler.

de nos concitoyens expatriés. L'article 2 de notre Constitution affirme : « La langue de la République est le français. » Mais comment s'assurer que tous les Français parlent la langue de la République, dès lors que, de plus en plus, les nouvelles générations qui naissent à l'étranger ne pratiquent pas le français ?

seul un jeune Français sur cinq à l'étranger suit l'enseignement offert par le réseau AEFE, cet amendement vise à réorienter une partie du budget vers les 80 % d'enfants français à l'étranger qui ne reçoivent aucune aide

Ce chèque éducation unique pourrait être utilisé exclusivement pour financer un enseignement du français ou en français, au sein d'un établissement du réseau AEFE,

le CIEP, pour s'assurer de la maîtrise du français acquise. La création de ce dispositif nécessiterait de transférer 30 millions d'euros du programme 151 vers le programme 185, notamment son action n° 02, Coopération culturelle et promotion du français. L'attribution de ce chèque éducation et son suivi seraient confiés à l'Institut français, dont la mission est justement d'assurer la promotion de la langue française en s'appuyant sur un réseau d'alliances françaises et d'instituts français bien plus développé et décentralisé que celui de l'AEFE, et qui permet donc de toucher davantage de familles. Quel

J'aurais aimé que tout le monde se rassemble autour de cet objectif : que tous les Français puissent apprendre à parler français ! Pour l'heure, je retire l'amendement.

l'initiative des représentants des Français établis hors de France, le dispositif « Français langue maternelle », ou FLAM, vise à soutenir des associations qui proposent à des enfants français établis à l'étranger, dans un contexte extrascolaire, des activités permettant de conserver la pratique du français en tant que langue maternelle et le contact avec les cultures française et francophones. Les associations peuvent ainsi bénéficier de subventions d'appui au fonctionnement au démarrage de leur projet, ainsi que de subventions pour l'organisation de regroupements régionaux d'associations FLAM.

et à en transférer la gestion à l'Institut français, dont la mission est justement d'assurer la promotion de la langue française, en s'appuyant sur un réseau d'alliances françaises et d'instituts français, qui, je le répète, est bien plus développé et décentralisé que celui de l'AEFE. Vous

Le doublement de ces crédits résulte de la conviction que l'apprentissage ainsi que la promotion de la langue française et du plurilinguisme constituent une nécessité et un atout dans la mondialisation, de même qu'un facteur de diversité indispensable. Cette mesure permettrait d'augmenter les dotations aux instituts français et les subventions aux alliances françaises, qui en ont besoin pour être de véritables acteurs de la modernisation de l'offre éducative et de la coopération linguistique.

dans la mondialisation, de même qu'un facteur de diversité indispensable, et ce dans tous les domaines : instituts français, subventions aux alliances françaises, etc. Quel est l'avis de la commission ?

plafonds empêchent nos instituts de disposer des moyens, c'est-à-dire des personnels, leur permettant de développer leur activité. C'est la raison pour laquelle la question des plafonds d'emplois mérite d'être posée dans cette discussion budgétaire. Quel est l'avis de la commission ?

Sur le fond, les frais de scolarité dont je parle n'ont rien à voir avec les frais de scolarité d'un établissement privé sous contrat en France. On évalue ces frais entre 4 000 et 15 000 euros par enfant. 4 000 et 15 000 euros par enfant. Chaque famille qui scolarise ses enfants participe au financement d'un établissement scolaire et au rayonnement de la France. Et ce n'est pas

en août 2018, de ne plus participer aux comités de prêts, qui aidaient à la préparation des dossiers de demande de garantie de l'État. Compte tenu de l'évolution du nombre des dossiers, de leur montant et des risques encourus,